vous avez déclaré que votre seule boussole était l'intérêt du justiciable et l'intérêt général. Je crains que vous n'ayez égaré la boussole En effet, nous avons appris l'existence d'un document, issu de votre cabinet, qui met scandaleusement en cause la neutralité du service public dont vous avez la charge. Madame le garde des sceaux, étiez-vous au courant de l'existence de ce document ? Deuxièmement, avez-vous demandé qu'il soit établi ? Troisièmement, puisqu'il a été communiqué au cabinet du Premier ministre, avez-vous reçu du Premier ministre

à l'égard de ceux qui sont responsables de cette atteinte intolérable à la neutralité du service public

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un vocabulaire simpliste et le portrait d'un chien, le président Trump a annoncé la mort du calife autoproclamé d'une organisation terroriste. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour devenir calife à la place du calife Le caractère nébuleux de ces organisations n'est plus à démontrer, et le chemin sera encore long avant que nous ne venions à bout de l'hydre terroriste. Les djihadistes ont certes beaucoup reculé et subi, ces derniers temps, des revers. Le groupe terroriste qui contrôlait la zone entre l'Irak et la Syrie a perdu beaucoup de terrain. Nombre de ses membres sont morts ou emprisonnés. Beaucoup de djihadistes occidentaux, notamment français, sont détenus dans des zones de troubles. Ne parvenant pas à trouver une solution qui soit satisfaisante, le Gouvernement a fait le choix de les laisser à leurs geôliers étrangers. Beaucoup d'entre eux risquent de parvenir à s'échapper, et ceux qui sont entrés dans la clandestinité pourraient revenir en France dans les mois qui viennent. À l'heure où l'Afghanistan est susceptible de redevenir une base arrière du djihadisme, à l'heure où le contrôle du Kurdistan syrien et des terroristes qui y sont détenus est fragilisé par une offensive unilatérale de la Turquie, il est à craindre que le risque terroriste n'ait pas pour autant disparu, notamment pour nos concitoyens, dans notre pays. Nous avons tous besoin de savoir à quelles menaces la France est aujourd'hui exposée du fait de cette situation. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, quel est l'état du risque terroriste en France et si de nouvelles mesures sont prévues pour les prévenir ?

chaque jour, à chaque instant, sur le territoire national, avec un risque terroriste élevé. Nous l'avons vu, hélas, ces dernières années, depuis 2015, avec les attentats terroristes, et même depuis 2013, lorsque les premiers ressortissants français se sont rendus sur les théâtres de guerre que vous évoquiez à l'instant, j'y reviendrai. Nous l'avons vécu récemment à Trèbes, à Strasbourg ou, plus récemment encore, à la préfecture de police de Paris, avec la mort de nombre de nos compatriotes. Oui, l'on voit combien nous devons vivre avec ce risque.

qu'il existe encore. Vous avez évoqué l'intervention américaine, qui a permis de neutraliser le chef terroriste dont je ne souhaite même pas prononcer le nom. J'ai immédiatement donné des instructions précises à l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure pour prévenir, au cas où, les risques de rebond ou de vengeance auxquels nous pourrions être confrontés. Je vous signale d'ailleurs que Daech n'a toujours pas reconnu, au moment où je vous parle, la neutralisation de celui qui fut son chef. Je n'exclus pas que le risque puisse être lié à ce moment d'expression. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de nos services de sécurité intérieure sont mobilisés en vue de parer les coups qui pourraient venir.

Ils sont systématiquement interpellés, judiciarisés et sanctionnés. C'est ainsi que nous continuerons de procéder pour tous ceux qui pourraient revenir du théâtre de guerre.

tout, de la cohérence gouvernementale, dont le Premier ministre a normalement la responsabilité. Mme Sylviane Agacinski a été privée par la présidente de l'université Bordeaux-Montaigne du droit de s'exprimer. Ce sont les faits. La réaction gouvernementale est surprenante. Mme Marlène Schiappa a sauvé l'honneur du Gouvernement en exprimant publiquement son désaccord. Qu'il en soit donné acte Mme le ministre de l'enseignement supérieur, qui est directement concernée, puisqu'il s'agit de l'université, a répondu d'une façon assez ambiguë à notre excellent collègue, Charles de la Verpillière, juriste éminent, qu'un forum serait organisé ... Je souhaite pour elle que ce forum soit accepté par les minorités qui avaient précédemment refusé l'intervention

vous ne respectez le droit de parler que si, et seulement si, les minorités turbulentes en donnent l'autorisation

des savoirs qui permette de penser ensemble notre monde et ses enjeux ». Que se passe-t-il donc à l'université ? Cette dernière manifestation a été annulée en raison, je cite les organisateurs, de « menaces violentes » émanant de « groupes » opposés aux positions de la philosophe sur les sujets actuellement en débat de la PMA et de la GPA, un débat qui viendra bientôt au Sénat et pour lequel, en amont, sont auditionnés tous les points de vue, ce qui reste encore l'une des meilleures façons de se construire un jugement. Comment en sommes-nous arrivés là ? Ces faits sont choquants pour nombre de nos concitoyens, car ils s'apparentent à des prises d'otages par des activistes identifiés qui font désormais ainsi régner, ici et là, une forme de terreur intellectuelle. Monsieur le ministre, mes questions sont assez précises : trouvez-vous normal que les présidents d'université concernés, sans doute eux-mêmes menacés, aient été obligés de céder aux injonctions de ces individus ? Pourriez-vous aussi nous dire, par conséquent, les mesures très concrètes que vous comptez prendre pour garantir au sein de ces établissements la liberté d'expression et les conditions de débats d'idées sereins ?

prolonger ma réponse. Tout comme vous, Frédérique Vidal et l'ensemble des membres du Gouvernement manifestent leur désapprobation de ce type d'actions extrémistes, qui vont contre la liberté de conscience et contre la liberté d'expression. C'est tout à fait contraire à toutes les traditions universitaires.

et nous ne l'accepterons pas

Le 16 octobre dernier, à la suite d'un accident survenu entre un TER et un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau dans les Ardennes, des centaines de conducteurs de train ont fait valoir leur droit de retrait, en solidarité avec le conducteur blessé, qui était seul à bord de son train. Depuis lundi, deux cents cheminots du technicentre de Châtillon ont également cessé le travail pour protester contre la remise en cause de douze journées de repos compensatoires, projet qui a été retiré La méthode a été contestée, car ce mouvement social inopiné, qui a commencé en pleine période de vacances scolaires, provoque d'importantes perturbations et la colère de millions d'usagers.

Ces actions semblent s'installer dans la durée et traduisent, à n'en point douter, un malaise chez les cheminots, qui est lié à des changements imminents et annoncés de direction et de statut, auxquels s'ajoute la prochaine réforme des retraites. Comment sont accompagnés ces changements à venir et, en particulier, celui du statut, qui interviendra le 1 janvier 2020 ? Monsieur le secrétaire d'État, je connais votre engagement en faveur du service public. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures sont prises pour un dialogue social de qualité ? La parole

vous l'avez dit, la SNCF connaît des transformations profondes : transformation de l'entreprise elle-même, le 1 janvier prochain, évolution des métiers, ouverture à la concurrence. Ces transformations peuvent être source d'inquiétudes pour les cheminots.

Il revient à celle-ci- le Premier ministre a été clair sur ce point -de prendre les mesures qui s'imposent envers les agents qui n'auraient pas respecté le cadre fixé par la loi. S'agissant du technicentre de Châtillon, le motif même de la grève est aujourd'hui invalidé, dans la mesure où le projet de réorganisation a été retiré par la directrice régionale. Dès lors, les demandes de primes n'ont pas de justification, et les jours de grève ne seront pas payés. C'est en tout cas la position réitérée de l'entreprise comme du Gouvernement.

Monsieur le ministre, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable interrogera la semaine prochaine le candidat aux fonctions de directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Yves Le Breton, déjà nommé commissaire général à l'égalité des territoires et chargé, à ce titre, de la préfiguration de cette agence. Auteurs de la proposition de loi qui a conduit à la création de l'ANCT, les membres de mon groupe s'intéressent bien sûr à son lancement et veilleront à ce que l'esprit initial du texte soit bien préservé.

; elle doit constituer un guichet unique à la disposition d'élus locaux aujourd'hui déstabilisés par la multiplicité des opérateurs et la complexité des procédures. Il était question non pas d'ajouter une strate supplémentaire au mille-feuille que tous les élus dénoncent, mais de leur simplifier la vie et de favoriser l'émergence de projets, grâce à un soutien accru en matière d'ingénierie, notamment dans les communes les moins dotées en moyens humains et financiers. Nous avons construit cette proposition de loi pour répondre aux attentes des territoires, qui aspirent à un service public pleinement utile, accessible et efficace.

Les deux questions sont directement liées, puisque, sans accès direct des élus locaux à l'ANCT, la raison d'être de cette dernière est clairement remise en cause. Par ailleurs, la publication du décret fixant la composition du conseil d'administration de cette agence devait intervenir avant le Congrès des maires, mais elle semble avoir été reportée. des territoires, a déjà répondu à de nombreuses questions sur ces sujets, mais les incertitudes demeurent ; il est urgent de les lever. Aussi, monsieur le ministre, j'aimerais que vous précisiez les missions de l'ANCT : est-elle destinée à décliner sur les territoires les programmes gouvernementaux ou, comme nous le souhaitons, à soutenir les projets des communes les plus fragiles ? Dans quelles conditions les élus locaux pourront-ils solliciter l'aide de l'ANCT ? Enfin, quelle place leur sera réservée au sein du conseil d'administration ? La parole

qui assurait, jusqu'à il y a peu, le transport de 400 000 tonnes de fruits et légumes entre Perpignan et le marché d'intérêt national de Rungis. Pourtant, le train a disparu ! Vous nous parlez d'urgence écologique, mais vous remettez sur la route 25 000 camions par an avec cette suppression Vous nous parlez d'amélioration de la sécurité routière et de la santé de la population, mais vous alimentez encore la surcharge des trajets domicile-travail avec ces véhicules additionnels et vous provoquez l'augmentation des nuisances, du stress, des ralentissements, de la pollution et des risques d'accident Grâce aux mobilisations, notamment celle d'élus qui sont présents aujourd'hui dans cet hémicycle et dont je tiens à saluer l'action, un comité de pilotage a été tardivement, mais finalement, mis sur pied, qui regroupe tous les acteurs concernés. Mes chers collègues, plus de quinze rencontres et visioconférences se sont tenues depuis mars 2019. Des élus, des acteurs économiques, des cheminotes et des cheminots, des citoyennes et des citoyens se sont mobilisés pour conserver ce mode de transport, le plus efficace économiquement et le plus écologique. Monsieur le secrétaire d'État, vous engagez-vous, oui ou non, à ce que cette ligne soit rouverte dès le mois de novembre 2019 ?

Voilà une semaine que des révélations concernant un e-mail adressé par votre ministère au cabinet du Premier ministre plongent le monde judiciaire et les élus dans le désarroi et la consternation. Ce document, destiné à élaborer une stratégie à adopter pour la suppression de certains cabinets d'instruction, des cibles et à opérer un tri en fonction des scores obtenus par le parti présidentiel et de la couleur politique des élus des municipalités concernées. Les villes potentiellement visées par ladite réforme se transforment en effet en véritables cibles électorales. Ce procédé est profondément choquant. Comment voulez-vous justifier, dans l'organisation territoriale de notre justice, une sanction envers les territoires qui ne voteraient pas comme il faut ? L'intrusion de considérations politiciennes dans l'ordre judiciaire est un manquement grave à la stricte séparation des pouvoirs et aux fondements de la démocratie.

et elle est simple ; j'espère donc obtenir de vous une réponse. Pouvez-vous nous assurer de la mise en place d'une procédure parfaitement transparente, avec des critères réellement objectifs, pour le regroupement territorial des pôles de l'instruction ?

sont pondérés par la prise en compte d'une réalité géographique- les distances entre territoires -, d'une réalité socio-économique

composés de magistrats, d'avocats et d'élus, seront systématiquement consultés. C'est écrit dans le texte de la loi ! Aujourd'hui, nous en sommes à des études préliminaires. Il est évident que ce processus est en cours.

Madame la garde des sceaux, même si vous tentez de minimiser la portée réelle de cette affaire, vos éléments de réponse n'apaisent en rien le profond malaise qui secoue la magistrature et les territoires. En effet, vos critères, madame la garde des sceaux, sont bien des critères politiciens,

le Sénat vous a soutenu, car nous vous faisions confiance pour agir dans l'intérêt du justiciable. En agissant de façon partisane, vous avez trahi cette confiance. Démission ! C'est aussi pour cette raison que notre commission des finances, lors de sa réunion d'hier, a décidé de ne pas approuver ces crédits pour 2020. Aujourd'hui, c'est avec une certaine amertume que nous constatons que ce lien de confiance est rompu par une politisation déplacée et indigne de la justice du XXI siècle.

une victoire pour nous tous, car nous nous étions tous fortement mobilisés contre cette coupe budgétaire inopérante et incohérente, qui portait gravement atteinte au monde agricole, mais aussi forestier. Nous avons été entendus : c'est bien, mais c'est insuffisant. Les inquiétudes demeurent ancrées : nous craignons de voir réapparaître un tel dispositif lors de la conclusion des contrats d'objectifs. Les chambres d'agriculture travaillent à l'accompagnement des professionnels

Non seulement le ruissellement annoncé n'a pas permis de revaloriser le revenu des agriculteurs, mais il a même pénalisé des PME alimentaires. La situation a empiré dans l'hyper-ruralité, notamment dans les zones défavorisées simples, où la réforme de agricole commune, a laissé sur le carreau de nombreux territoires, comme la Piège, dans l'Aude, ou encore le Gers. Et que dire des inquiétudes grandissantes sur l'avenir de notre PAC ? Chiffre effarant, un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 euros par mois ! Comment peut-on, au XXI siècle, assurer le renouvellement des générations dans l'agriculture quand la promesse de revenus à venir est insuffisante ? C'est un défi immense pour la France, qui va voir un tiers de ses exploitants partir à la retraite avant 2030- et quelle retraite ! Aussi, ma question est la suivante que dites-vous aux paysans qui ont tant espéré du ruissellement promis par la loi Égalim et pour qui le compte n'y est pas ? Concrètement, comment allez-vous contraindre la grande distribution à mieux répartir la valeur ? La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Nous avons souhaité encourager, au travers de la mesure que vous avez évoquée, la modernisation du réseau des chambres d'agriculture, ce que ces dernières reconnaissent volontiers. C'est dans ce contexte que nous avons proposé de diminuer de 45 millions d'euros le produit de la taxe affectée. Après un dialogue approfondi avec l'ensemble des parlementaires, y compris les sénateurs, le Gouvernement a décidé de retirer cette mesure du projet de loi de finances, afin d'engager une plus large concertation, qui prenne notamment en compte les questions de péréquation entre chambres d'agriculture et la question de la filière bois.

construction des prix devait se faire sur la base du coût de production. Un an après le vote de la loi Égalim, il appartient aujourd'hui non seulement au Gouvernement, mais aussi à l'ensemble des acteurs du monde de l'agriculture, de peser pour observer la construction des prix et vérifier que les termes de la loi sont bien respectés. Un an après, on constate des avancées dans un certain nombre de secteurs ; je pense à la filière lait ou à la filière porc. Reconnaissons cependant-

vous travaillez depuis deux ans à une réforme des retraites et, la semaine dernière encore, vous avez été désavoué par le Président de la République quant au modèle que vous proposiez. Vous aviez annoncé un aboutissement de la réforme avant les municipales, puis après les municipales- ce qui est plus sage ! Cela semble maintenant repoussé aux calendes grecques. Vous nous avez proposé de passer d'un système par répartition à un système par points. Vous avez annoncé la fin des régimes spéciaux, mais on apprend par la presse que cela tangue au sein du Gouvernement. Vous avez vous-même affirmé que l'option d'une réforme des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants n'était pas votre tasse de thé Président de la République. En vérité, une seule chose semble sûre : vous avez fait le choix de la baisse du pouvoir d'achat des retraités, puisque les pensions ne seront pas revalorisées en 2020. le temps est venu de tomber les masques, de regarder les Français dans les yeux et de leur dire la vérité, sans « en même temps » permanent, sans en même temps et en permanence ménager la chèvre et le chou. Peut-être craignez-vous de revivre les grèves de 1995 ... Je vous poserai deux questions. Premièrement, êtes-vous prêt à proposer la suppression immédiate des régimes spéciaux et l'alignement des régimes du public sur ceux du privé sans décaler la réforme, quitte à introduire un peu de progressivité ? Deuxièmement, êtes-vous prêt à reconnaître que notre système par répartition ne peut être maintenu que s'il y a un allongement de la durée de cotisation, du fait de l'espérance de vie qui s'allonge et du ratio entre bénéficiaires et cotisants, aide, monsieur le ministre.

mettre en place un système universel des retraites, avec des principes extrêmement clairs : mêmes règles pour tous ; à carrières identiques, cotisations identiques et retraites identiques ; mise en place d'un régime universel, dont le but est de supprimer la totalité des régimes spéciaux-

La seule chose qui apparaisse évidente, c'est que les pensions vont baisser en 2020, puisque c'est inscrit dans le projet de loi de finances. Le véritable courage aurait sans doute été d'admettre que, pour maintenir le niveau des pensions, il faut augmenter le temps de cotisation, comme l'ont fait d'ailleurs tous les pays voisins. Le Président de la République affirme qu'il veut aller jusqu'au bout de cette réforme ... Mais de quelle réforme s'agit-il ?

Cela s'applique dès le 1janvier 2020, à la suite d'un décret du mois de juillet dernier. Dans la vraie vie des blocs, à deux mois de l'échéance, où en est-on ? Actuellement, ce sont des infirmiers diplômés d'État qui font fonction d'Ibode, et l'on estime qu'ils sont majoritaires dans un grand nombre de blocs. Sans eux, pas de chirurgie. Depuis 2015, les objectifs de formation sont très loin des besoins, malgré une augmentation légère des inscriptions : de 390 en 2016, celles-ci sont

chère, chronophage. Très peu d'infirmiers ont choisi cette voie, alors qu'ils sont pourtant nombreux à en avoir largement les compétences. Sur ces sujets se greffent les questions de statut et de valorisation salariale peu attractives et non encore réglées. Vous le savez, madame la secrétaire d'État, il y a urgence. Si les conditions d'accès au diplôme qualifiant, le calendrier et la faible reconnaissance statutaire sont maintenus en l'état, c'est la paralysie de l'activité chirurgicale qui s'annonce durablement. C'est bien sûr inenvisageable : ni les patients, ni l'hôpital, ni les praticiens ne doivent subir les effets de ce noeud administratif anxiogène. Aussi, madame la secrétaire d'État, je vous demande quelle solution vous comptez apporter pour pallier en urgence cette situation.

de la santé. Madame la sénatrice, sachez que nous partageons votre préoccupation d'assurer la pérennité de l'activité opératoire, en France. La question que vous posez est précise, et la réponse le sera tout d'autant. Le décret du 27 janvier 2015 attribue aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, les Ibode, de nouveaux actes qualifiés d'exclusifs, que vous avez rappelés : aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration au cours d'une intervention chirurgicale en présence du chirurgien. suite d'un recours, le Conseil d'État a différé l'entrée en vigueur de ces trois actes exclusifs, et un dispositif transitoire a dû être mis en place. Ce dernier permet de garantir la compétence des professionnels autorisés à réaliser les trois actes concernés sans compromettre la continuité des activités opératoires. Ce dispositif transitoire, mis en oeuvre jusqu'en 2021, consiste à satisfaire à une épreuve de vérification des connaissances devant une commission régionale. Tout en préservant le principe de l'exclusivité des infirmiers diplômés d'État de bloc opératoire, ce dispositif transitoire maintient la possibilité pour les infirmiers expérimentés, à titre dérogatoire, de continuer à réaliser ces actes au regard de leurs compétences et de préserver la sécurité et la continuité des soins. Au-delà de ce sujet, les travaux sont d'ores et déjà programmés dès le mois prochain, avec l'ensemble des partenaires- employeurs et représentants des infirmiers de bloc -, concernant la question de la démographie de la profession et au cours desquels sera aussi traitée la question de l'attractivité de ces métiers. La parole

aussi une problématique de financement. La santé a un coût, la population vieillit, les moyens thérapeutiques et les diagnostics sont de plus en plus chers. Il faudra que nous l'assumions tous, collectivement. J'espère et j'attends de votre gouvernement qu'il l'assume aussi et qu'il l'affirme. La parole

recensant les mauvais résultats de la France en matière d'émissions de CO2, de dégradation de la biodiversité ou de qualité des eaux souterraines. Ces faiblesses chroniques en matière environnementale sont à rapprocher de l'échec violent de votre politique fiscale, privilégiant une écologie punitive, ayant mis le pays en très grande tension l'an passé, à la suite d'une hausse brutale, non concertée et confiscatoire de la taxe carbone. Dans le contexte de changement climatique actuel, sur la base de ces mauvais résultats, alors même que, en un peu plus de deux ans, trois ministres ont déjà été en charge de l'écologie, allez-vous mener une politique disruptive ou bien mettre vos pas dans ceux de MM. Hulot et de Rugy ?

en déplacement. Le Gouvernement a pris acte de l'arrêt du 24 octobre dernier de la Cour de justice de l'Union européenne relatif au non-respect des normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote. Vous n'êtes pas sans savoir que ce problème ne date pas d'hier. Je rappelle par ailleurs que, sur la période 2000-2018, les émissions d'oxyde d'azote ont baissé de 54 % et que le nombre d'agglomérations concernées par les déplacements de la valeur limite a été diminué de moitié. Cela n'est pas suffisant, et je veux vous assurer de la totale mobilisation du Gouvernement sur le sujet. Cela passe par une série de mesures structurantes déjà engagées, telles que l'accompagnement au renouvellement du parc automobile, le développement de bornes électriques, l'aide aux particuliers pour renouveler les appareils de chauffage, ou encore l'accompagnement financier des collectivités, au travers des dispositifs de l'Agence De nouvelles actions sont inscrites, notamment dans la loi d'orientation des mobilités, dont nous avons eu à débattre ces derniers mois. Ces actions portent sur le déploiement des zones à faible émission dans les métropoles, qui sera obligatoire dès lors que les collectivités dépassent régulièrement les valeurs limites. Elles passent aussi par la mise en oeuvre du plan Vélo qui, comme vous le savez, triplera d'ici à 2024 la part des déplacements du vélo dans les transports du quotidien. Elles passent encore par la création du forfait mobilité durable visant à inciter les employés à utiliser le vélo ou le covoiturage pour leurs trajets du quotidien, ou encore par la réduction des émissions des navires à quai au travers du plan Escales zéro fumée. Monsieur le sénateur, c'est bien ce gouvernement qui a proposé la mise en oeuvre de ces mesures pour apporter une solution aux conséquences dramatiques de la pollution de l'air. au mois de juillet dernier, vous avez décidé, six mois après avoir décidé la prime à la conversion, de changer les règles. Honnêtement, cela ne se fait pas ! En outre, alors que vient d'être adoptée la loi d'orientation sur les mobilités, vous ne permettez pas aux intercommunalités de conduire leur politique En ce qui concerne le crédit d'impôt de transition énergétique, vous venez de sortir pratiquement la moitié des Français du dispositif d'aide et de soutien, alors qu'il faut aujourd'hui examiner la réussite de l'étiquette énergétique. Nos paysans

Madame la secrétaire d'État, en France, de 8 à 11 millions de personnes soutiennent un proche en perte d'autonomie, soit un Français sur

Qu'est-ce qu'être un aidant ? C'est Claude qui accompagne sa mère dans son quotidien, de la préparation des repas aux tâches administratives, aux sorties, à la toilette. C'est ce père qui a demandé à son employeur de passer à temps partiel pour s'occuper de son fils, Enzo, handicapé à 85 %. L'amour et le dévouement qu'ils portent à leurs proches sont inconditionnels il n'en demeure pas moins qu'ils sacrifient souvent une carrière, une retraite, voire une vie sociale. Madame la secrétaire d'État, vous êtes une mère concernée par le handicap et une militante associative de longue date. Votre investissement sur ce sujet n'est plus à démontrer. Aux côtés de M. le Premier ministre et avec le concours des représentants des proches aidants, vous avez eu à coeur d'élaborer une stratégie de mobilisation et de soutien en leur faveur. Cette stratégie, qui incarne l'ambition d'une société plus attentive et solidaire, se traduit dans le principe par un financement sur trois ans, à hauteur de 400 millions d'euros, par un déploiement des mesures à partir de 2020 et par un comité de suivi deux fois par an. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous détailler les mesures qui permettront, d'une part, d'améliorer la qualité de vie des aidants, et, d'autre part, de reconnaître leur rôle pour une société plus solidaire et adaptée à la perspective d'une forte hausse de la perte d'autonomie ? La parole

Une étape très importante a été franchie avec la reconnaissance des proches aidants dans nos politiques publiques, y compris lorsqu'ils sont très jeunes- plus de 500 000 d'entre eux le sont -, dans -, dans le prolongement d'un travail parlementaire, auquel le Sénat a beaucoup contribué et qui a ouvert la voie, ainsi que d'un travail associatif très important, que je tiens à saluer.

un congé proche aidant rémunéré de trois mois beaucoup plus accessible, fractionnable, sans condition d'ancienneté- voilà qui résoudra les problèmes de Claude aujourd'hui -, la défiscalisation du dédommagement versé à l'aidant familial, dans le cadre de la le soutien au répit avec des plateformes régionales qui pourront donner des réponses graduées, par exemple le relayage- un accompagnant vient vous remplacer pour vous permettre de prendre des vacances -, de l'accueil temporaire, des solutions de vacances adaptées. Voilà, monsieur le sénateur, des mesures qui seront applicables dès 2020. Je me réjouis que nous puissions travailler tous ensemble sur ce sujet. Je pense que nous devons être solidaires envers ceux qui le sont déjà. La parole

Vous l'avez tellement bien compris que vous renvoyez désormais aux présidents des départements la responsabilité d'une décision non concertée, qu'ils n'ont jamais souhaitée. Ils vous avaient pourtant mis en garde.

différentes d'un département à l'autre. Ce ne sera pas un gage de lisibilité et de sécurité pour les automobilistes. Aussi, monsieur le Premier ministre, mettez fin à cette hypocrisie, à cette « guéguerre » des experts, chiffres contre chiffres. Faites cesser ces querelles stériles, qui fracturent nos territoires ! Vous seul pouvez le décider. Revenez sur votre décret du 15 juin 2018. Revenez aux 90 kilomètres par heure. Les élus sauront prendre leurs responsabilités.

mais, attention, ce n'est pas parce que vous affirmez quelque chose que c'est une vérité. Vous non plus ! Ce n'est pas parce que j'affirme quelque chose que c'est une vérité. Il faut, monsieur le sénateur, écouter, et non pas stigmatiser, en particulier le Conseil national de sécurité routière.

La politique économique menée depuis 2017 fait-elle augmenter le nombre de pauvres ? » s'est interrogée la presse. Tel autre journal a titré : « Misère et inégalités s'accentuent », selon l'Insee, Ainsi, près de 15 % de la population auraient des revenus inférieurs au seuil de pauvreté, ce qui signifie que plus de 9 millions de personnes vivent avec moins de 1 050 euros par mois. Derrière ces chiffres, il y a une réalité dramatique : c'est la mère qui ne peut donner à manger à ses enfants,

détenteurs d'actions. Ces ménages ont aussi bénéficié de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, qui abaisse la fiscalité sur ce type de revenus, moins imposés que les revenus du travail. Il est à noter que ces données provisoires ne prennent pas en compte la réforme de l'impôt de solidarité

n'est pas à la hauteur des enjeux sociaux, c'est deux fois moins que les cadeaux fiscaux aux plus riches ... ». Bref, il est plus que temps de changer de dimension.

de la prime d'activité, au reste à charge zéro, à la nouvelle complémentaire santé solidaire, qui s'adresse aux personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, qui vont pouvoir bénéficier d'une couverture

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis que le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la France a un passé industriel et, surtout, un avenir industriel. C'est pour cette raison que le Sénat s'est attaché depuis plusieurs années à travailler sur le sujet de l'industrie. Il y a déjà près d'un an et demi, la mission d'information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays rendait ses conclusions. Alors que les temps sont aujourd'hui aux start-up et au numérique post-industriel, il n'en est pas moins nécessaire de conserver une industrie forte et modernisée, car la production métallurgique, notamment, constitue un enjeu essentiel pour notre économie et son autonomie. L'acier se trouve au sommet de la chaîne de valeur de nombreuses industries. Sa production nécessite des investissements importants, avec des seuils de rentabilité élevés et des marges faibles. L'acier est pourtant un enjeu de souveraineté. Il forge nos armes, au sens propre. Les vecteurs de notre force nucléaire- avions et sous-marins principalement -nécessitent des alliages spéciaux en acier de haute technicité. L'acier est aussi un enjeu pour la transition énergétique. Le recyclage de l'acier représente une contribution importante dans le cadre de notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier les évolutions technologiques qui permettent de limiter les émissions de CO2 dans la filière chaude au sein des hauts-fourneaux. Or, douze ans après le Grenelle de l'environnement, la politique de l'éco-conception reste trop virtuelle et l'éco-recyclabilité des produits industriels à base d'acier est encore trop peu développée. La France et l'Europe sont devenues des acteurs marginaux sur le marché mondial de l'acier, aujourd'hui dominé par la Chine, qui représente 50 % de la production mondiale. Seuls les trois quarts à peine des capacités de production existantes sont utilisées. Nous sommes aujourd'hui en pleine crise de surcapacité, la création de nouvelles capacités se poursuivant dans un contexte de guerre commerciale exacerbée entre la Chine et les États-Unis. Pourtant, malgré les efforts de structuration de la filière, il nous manque une politique publique claire, un ministre de l'industrie et des moyens humains et financiers dédiés. manque également une véritable vision industrielle européenne. En effet, l'Europe est aujourd'hui trop focalisée sur la politique de concurrence, ce qui a pour conséquence première d'entraver notre capacité à construire des géants économiques capables d'affronter la concurrence mondiale. Le dossier Alstom-Siemens en est un exemple. Enfin, l'Europe est trop lente à réagir face au dumping et elle manque d'ambition industrielle. Nous avons besoin d'une Europe stratège pour notre industrie. Dans ce contexte, la mission d'information que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider a, pendant cinq mois, entendu 55 personnes et effectué plusieurs déplacements sur le terrain. J'en profite pour remercier mes collègues membres de la mission,

à l'heure où la réindustrialisation des territoires est un objectif partagé du Gouvernement et des élus locaux, la consolidation de notre industrie sidérurgique nationale est absolument stratégique. Notre mission d'information a identifié trois défis majeurs pour le futur de la sidérurgie française. Tout d'abord, la surcapacité de production persiste à l'échelon mondial, exacerbant la concurrence, au détriment de l'industrie européenne. De plus en plus de pays, en particulier la Chine, ont recours au protectionnisme commercial et à des pratiques déloyales. Ensuite, les sidérurgistes doivent prendre le virage de la transition énergétique. L'acier doit nécessairement devenir plus vert, mais les objectifs climatiques et énergétiques se renforcent et la hausse du coût du carbone s'accélère sur le marché des quotas, alors que les pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Enfin, les moyens nécessaires à l'adaptation de l'industrie sidérurgique sont difficiles à mobiliser, alors que les investissements sont particulièrement lourds

Pour donner des armes à l'acier français dans la compétition mondiale, nous avons formulé trente recommandations, qui agissent sur quatre leviers. Le premier est le soutien de la transition énergétique à la sidérurgie française. Alors que le prix de la tonne de carbone à l'échelon européen augmente depuis quelques mois, il serait inacceptable que ce renchérissement renforce la compétitivité des entreprises situées en dehors de l'Union européenne et qui ne sont pas soumises aux mêmes contraintes, alors même que leurs émissions de CO2

les investissements des entreprises sidérurgiques pour décarboner la filière ne porteront leurs fruits qu'à la condition d'être soutenus par un coût de l'énergie compétitif. La compétitivité du prix de l'énergie en Europe est un élément déterminant dans les choix d'investissement des groupes sidérurgiques et conditionne l'avenir de la filière. À l'échelon national, le coût de la compensation carbone, compensant les coûts des quotas carbone qui sont répercutés sur le prix de l'électricité pour des secteurs exposés à un risque de fuite carbone, est appelé à augmenter ces prochaines années.

Le second levier est la défense de nos intérêts commerciaux et la protection du marché sidérurgique européen contre des compétiteurs aux pratiques déloyales. L'industrie européenne utilise de plus en plus d'acier importé, au très mauvais bilan carbone et largement financé par des subventions des États. Pour restaurer des conditions équitables, il faut une politique volontariste de la Commission européenne, qui doit se saisir pleinement de ses nouveaux outils de défense commerciale, aujourd'hui insuffisants et plus adaptés. Il faut absolument les revisiter, à un rythme différent du tempo européen habituel. Le troisième levier est la stratégie de filière, qui améliore l'articulation entre les besoins des entreprises sidérurgiques et le soutien des pouvoirs publics. Il faut que les industriels s'impliquent fortement dans ces projets structurants, qui bénéficient à tous, et que l'État engage plus de moyens pour améliorer le dialogue. Le quatrième levier, le plus essentiel, c'est, comme l'a dit mon collègue Franck Menonville, l'accompagnement stratégique à tous les niveaux des politiques publiques. Pour mobiliser pleinement les trois autres leviers et renforcer le pilotage de la politique industrielle, il faut mettre en place un véritable ministère de l'industrie, pas symbolique, mais doté de moyens humains et budgétaires appropriés, ce qui n'est plus le cas depuis trop longtemps, madame la secrétaire d'État. Ce n'est pas le fait de ce gouvernement, mais ce gouvernement peut changer les choses et faire de la sidérurgie une véritable priorité nationale. Seul un tel- ou une telle ! -ministre de l'industrie

Il rassemblera tous les acteurs concernés autour de la table, en lien avec le Conseil national de l'industrie, dans une approche partenariale avec l'échelon territorial et régional, premier maillon de l'accompagnement des bassins sidérurgiques.

projet de loi de finances pour l'année 2020 ? Nous sommes à la croisée des chemins à l'échelon européen ; beaucoup de décisions vont être prises. Que comptez-vous faire ? La parole

monsieur le président de la mission d'information, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez raison, la sidérurgie est un maillon central de l'industrie française. L'importance de la sidérurgie est notamment liée à sa place incontournable dans de nombreuses filières industrielles majeures. C'est le cas en particulier de la construction,

emploient plusieurs milliers de salariés dans les bassins des Hauts-de-France, du Grand Est, des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sa présence est aussi le fait de nombreuses usines de plus petite taille, aciéries électriques ou unités de transformation aval- laminoirs, fonderies. C'est un secteur mondialisé, qui doit s'adapter à une concurrence féroce. Face à l'agressivité de la concurrence mondiale en termes de prix, de volumes, de capacités, de concentration, les acteurs de la filière ont su se transformer afin de rester dans la course : restructuration des aciers plats français, qui détiennent maintenant une bonne position de marché, transformation et sécurisation des emplois du site de Florange, où 2 200 emplois ont été conservés

et développement, la transformation numérique des entreprises, la sécurisation des approvisionnements en matières premières, l'attractivité de ses métiers. Tous sont importants, mais quelques-uns me semblent vitaux pour l'avenir de la filière sidérurgique française et européenne. Le premier enjeu est de traiter la surcapacité mondiale, ce qui renvoie à la proposition n° 6. En dix ans, la Chine est devenue le premier producteur mondial d'acier. À elle seule, elle produit 930 millions de tonnes d'acier, soit plus de 50 % de la production mondiale, et elle est responsable de la moitié des surcapacités mondiales qui pénalisent les aciéristes européens, tirent les prix à la baisse et détruisent les marges en Europe. Or les marges sont la condition des investissements et des emplois. Les aciers plats ont ainsi vu leur prix baisser de 21 % entre janvier 2018 et mai 2019. Sous l'impulsion de l'Union européenne et des États-Unis, le G20 a mis en place en 2016 un forum mondial sur les surcapacités dans le secteur de l'acier, le GFSEC.

8 et 27 de votre rapport. Près de la moitié des cas anti-dumping ou anti-subvention traités à l'échelon européen relèvent du seul secteur de la sidérurgie. Les règles de concurrence loyale ne sont en effet pas toujours respectées par nos partenaires. Vous le savez, nous poussons la Commission européenne à renforcer son action en la matière. C'est d'ailleurs ce que je fais au conseil Compétitivité. Le troisième enjeu est de faire de l'impératif climat une chance avec la proposition n° 9. Les enjeux climatiques sont aujourd'hui un impératif reconnu par tous. Le plan Climat du Gouvernement et sa déclinaison dans la stratégie nationale bas-carbone fixent l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. La sidérurgie est responsable d'environ 7 % des émissions anthropiques de CO2 dans le monde. À ce titre, elle a une responsabilité envers la planète, mais elle fait aussi face elle fait aussi face à d'exceptionnelles occasions de rupture technologique qui permettront aux industriels les plus offensifs de se différencier- j'y reviendrai. Le quatrième enjeu, celui de la compétitivité, passe par un engagement fort sur le prix de l'électricité ; cela renvoie aux propositions n 13 et 15.

les efforts actifs que nous avons réalisés pour défendre notre budget de compensation CO2. Je pense notamment à la réflexion que nous avons engagée pour faire en sorte que les entreprises intensives et les hyper électro-intensifs bénéficient,

Le crédit d'impôt recherche, que de nombreuses nations ont copié, est un outil souple et massif de soutien à la R&D des entreprises. En revanche, nous avons des marges de progrès s'agissant de l'industrialisation de la R&D sur le territoire national. Il faut y travailler tous ensemble. Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer en la matière. C'est notamment en offrant aux investisseurs

constant pour l'industrie, qui s'est renforcé cette dernière année. Depuis sa création, elle a été présente sur de nombreux dossiers du secteur des métaux. Elle a été associée à de grands succès, comme Constellium, auquel j'ai personnellement participé en 2009. elle est une actrice cruciale dans les dossiers plus sensibles, comme Vallourec. Bpifrance est un investisseur avisé en économie de marché soumis aux règles de concurrence communautaire en matière d'aides d'État. Elle n'intervient pas directement en retournement, mais elle gère pour le compte de l'État le Fonds de fonds de retournement, ou FFR, doté de 74,7 millions d'euros dans le cadre du programme d'investissements d'avenir, qui souscrit à des fonds gérés par des équipes spécialisées et dont nous avons besoin sur certains dossiers. Je tiens

Je me contenterai de rappeler, trois exemples concrets, que la stratégie industrielle de l'État s'est structurée et renforcée durant ces deux dernières années. La stratégie de filière a été renforcée. Le 18 janvier dernier, j'ai signé le contrat stratégique de filière Mines et métallurgie avec la présidente du comité stratégique de filière, Mme Christel Bories, en présence des organisations syndicales. C'est une instance unique, où tous les acteurs, entreprises, organisations syndicales et administrations peuvent échanger hors situation de crise pour consolider et préparer ensemble l'avenir de la filière. Ils travaillent ensemble sur plusieurs sujets importants soulevés dans le rapport : l'avenir des différentes filières acier en France- hauts-fourneaux et aciéries électriques -, la réduction des émissions carbone, la lutte contre la concurrence déloyale, la transformation numérique de la filière, la sécurisation des approvisionnements en matières premières, l'attractivité de ses métiers.

Le Gouvernement est très attentif à ce risque. À ce titre, et dans le cadre du Conseil national de l'industrie, le CNI, le Conseil général de l'économie a remis au ministère de l'économie un rapport sur la vulnérabilité de l'approvisionnement en matières premières des industries françaises, ce qui a permis d'identifier plusieurs pistes de travail. Pour les mettre en application, exécutif, le Comex, du CNI du 23 septembre dernier le lancement de travaux applicatifs sur la sécurisation des approvisionnements en matières premières associant des industriels de référence de l'amont, producteurs de métaux, et de l'aval, consommateurs, pour trois filières d'excellence et d'avenir fortement consommatrices de métaux critiques les batteries pour la mobilité, les énergies renouvelables et le secteur de l'aéronautique et défense. Les conclusions sont attendues pour la fin de l'année 2019, et des premières applications pratiques ont été mises en oeuvre. Des travaux sur l'avenir des aciéries électriques sont menés ; cette question est liée à la proposition n° 16. Je l'ai déjà souligné, la filière des hauts-fourneaux en France s'est restructurée et elle est maintenant au meilleur niveau européen et mondial. En revanche, les aciéries électriques françaises ont subi une succession de difficultés, que votre rapport a relevées et qui ont entraîné des fermetures de sites et des arrêts définitifs de fours. Pourtant, la filière électrique dispose de caractéristiques qui devraient lui permettre de soutenir un développement concurrentiel : plus faible intensité capitalistique que les hauts-fourneaux, flexibilité, adaptation aux aciers de spécialité et aux petits volumes, réactivité opérationnelle ... Par ailleurs, avec une faible émission de CO2 à la tonne, l'aciérie électrique est un élément de réponse à la réduction des émissions de la filière et à l'objectif de décarbonation de l'économie. Je me félicite donc que le comité stratégique de filière Mines et métallurgie vienne de lancer un groupe de travail pour dégager des scénarios de développement des différentes technologies de production de l'acier en France associant les industriels, les organisations syndicales et les administrations. C'est un travail fondamental, qui doit éclairer l'avenir. Ce type de travaux est dans l'ADN des comités stratégiques de filière et fait partie des réflexions stratégiques et de l'anticipation qui sont indispensables pour l'avenir de l'industrie et dont votre rapport souligne l'impérieuse nécessité.

un éclairage sur la situation. Madame la secrétaire d'État, je vous invite à conclure. J'aimerais mentionner une dernière action en matière de formation. C'est le principal défi de la filière. La filière est en tension. Elle peine à recruter et doit faire évoluer ses compétences pour s'adapter aux nouvelles donnes introduites notamment par la numérisation de l'économie.

La situation périlleuse de notre industrie sidérurgique est principalement la conséquence du développement exponentiel de la concurrence étrangère. En 2017, près de 1 700 millions de tonnes étaient produites à travers le monde, dont près de la moitié en Chine. Les trois principaux pays producteurs d'aciers, tous situés en Asie- il s'agit de la Chine, du Japon et de l'Inde -, totalisent plus de 68,8 % de la production mondiale. Pourtant, aujourd'hui, malgré plusieurs mesures anti-dumping mises en place pour renforcer la compétitivité de nos entreprises, la question reste en suspens : de l'avenir de l'acier français ? La richesse de notre industrie française se concentre aujourd'hui dans le développement de nouveaux savoir-faire. J'ai donc deux questions. La technologie La technologie peut être une issue pour notre industrie. En 2017, le sidérurgiste américain Nucor, qui représente 30 % de tout l'acier américain, avec dix-huit aciéries électriques, a aligné des performances de premier plan un recyclage massif, un souci de l'environnement, quatre fois moins de CO2 par tonne produite que ses concurrents et des dividendes redistribués durant 180 trimestres successifs depuis 1972. Comment accompagner nos entreprises dans la restructuration de leur modèle économique ? Par ailleurs, je pense que les préoccupations environnementales peuvent être une chance. L'acier présente quelques avantages pour le développement durable : filière sèche, faible consommation en eau, peu de déperditions énergétiques, longévité des matériaux et facilité dans la déconstruction, notamment par rapport au béton. L'acier peut même être à 100 % recyclable. Comment, là encore, accompagner nos entreprises sidérurgiques, pour en faire des acteurs du développement durable et de l'économie circulaire ?

la France est capable de proposer des solutions en la matière, elle pourra regagner des parts de marché et, en effet, augmenter sa compétitivité. Je tiens à le rappeler, la sidérurgie française est présente sur les aciers les plus modernes à valeur ajoutée à la fois par sa filière des hauts-fourneaux, avec des aciers techniques pour l'automobile, comme Usibor d'ArcelorMittal, par des aciéries électriques très haut de gamme sur les superalliages et les alliages de titane mis en oeuvre par Aubert et Duval, ainsi que par des inox et des produits très spécialisés, comme les aciers à grains orientés par les transformateurs. Vous mettez l'accent sur sur les choix de technologie du type aciérie électrique, sur lesquels on doit notamment tenir compte des investissements passés, de la base industrielle installée, des ressources et de l'évolution de la demande. La décarbonation de la production d'acier dans les hauts-fourneaux réduira à à terme très fortement leur émission. C'est une première réponse. De nombreux projets de R&D sont déjà engagés pour cela, car la filière fonte restera essentielle dans l'offre d'acier des prochaines années eu égard aux projections de la demande. La filière électrique est cependant une technologie moderne également majeure. Elle dispose de caractéristiques qui devraient lui permettre de soutenir un développement concurrentiel, une plus faible intensité capitalistique, la flexibilité, l'adaptation à cette spécialité. À court terme, elle est handicapée,

mêmes réponses. Et pendant ce temps, les sites industriels sont délocalisés, avec les emplois perdus et les ravages économiques et sociaux qui vont avec ! Aucun territoire et aucune filière n'ont été épargnés par les fermetures deux sites d'Ascométal dans la filière électrique ; chez Eramet, l'aciérie électrique de Firminy ; pour les cylindres, Akers, et Vallourec a fermé ses laminoirs de Saint-Saulve et de Déville-lès-Rouen ; dans la filière fonte, c'est l'arrêt de Florange. Entre 2013 et 2017, la sidérurgie a perdu près de 10 000 emplois directs. Autant de vies et de savoir-faire détruits au nom de la compétitivité. Une véritable hécatombe

soit il y a une volonté non assumée de sacrifier la sidérurgie et, par là même, notre tissu industriel, sur l'autel du profit. Si c'est cela, il faut le dire clairement Combien de temps allons-nous encore constater la faiblesse de l'État actionnaire face aux appétits capitalistes et l'absence de stratégie industrielle sur le long terme ? Est-ce Est-ce que votre politique industrielle se résume à voir nos outils industriels partir à l'étranger, à être naïfs dans la guerre économique, à subventionner les entreprises à hauteur de 200 milliards d'euros sans demander de contreparties en termes d'emplois et d'investissements en attendant que la « main invisible » du marché vide la France de son industrie ? Ou alors allez-vous enfin interdire les délocalisations de site dans les filières que nous considérons comme stratégiques et mener une politique industrielle audacieuse, en commençant par nommer un ministre de l'industrie ? La parole est à Mme la secrétaire

ou de l'emploi. Mais cette action se limite à présent presque exclusivement à la gestion de crise, pour éteindre des feux. Le dossier Ascoval montre bien à quel point même la gestion de crise est difficile. Le rapport de notre collègue fait ainsi état d'un enchaînement de mauvaises décisions et de déclarations précipitées, qui témoigne de l'absence de stratégie française en la matière. Il nous semble pourtant essentiel de mettre en place le cadre légal favorable au développement de l'industrie. Que peuvent faire nos industriels face à une taxe carbone qui, en Europe, ne s'applique pas aux importations ? L'émergence d'acteurs solides, capables de soutenir une concurrence mondiale face à d'autres grands acteurs, doit être encouragée. Nous avons vu, lorsque General Electric a racheté la branche énergie d'Alstom, que d'autres États soutiennent très activement leurs industriels. La France doit protéger son industrie et ses savoir-faire. Elle doit soutenir l'investissement dans les secteurs stratégiques. Mais, comme il n'y a plus ni ministre ni secrétaire d'État à l'industrie, comment pourrait-elle avoir une vision stratégique ? Une vision stratégique est indispensable. Elle dépasse aujourd'hui le cadre national. Elle doit être européenne. On ne pourra pas faire l'économie de l'adaptation aux règles de la concurrence, mais le sort de notre industrie se joue maintenant.

les innovations, la transition écologique énergétique et l'approvisionnement en métaux rares. Le dispositif Territoires d'industrie, qui est au plus près des territoires, en lien avec les collectivités locales, permet de défendre des projets, notamment pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire.

Tous ces éléments font une vision et une stratégie industrielles. Oui, nous prenons aussi le temps d'accompagner les entreprises en difficulté. C'est notre travail ! D'ailleurs, ce ne sont pas les dossiers les plus difficiles. Mais je veux vous rappeler ici

le cap ? Peut-on croire à un discours de vérité ? Je suis élue de la Nièvre. Sur le site Vallourec de Cosne-Cours-sur-Loire, les élus et les salariés ont fait les frais de ces évolutions spasmodiques. Nous avons tous eu l'impression de courir derrière des décisions dont la stratégie nous échappait.

Les cessions-reprises à suspense, qui apparaissent parfois comme des liquidations en plusieurs temps parfaitement orchestrées, ne peuvent pas nous faire croire que la transparence est revenue. Le directoire annonce que l'amélioration des performances du groupe se confirme et que le chiffre d'affaires annuel est en hausse ; je m'en félicite. Les tubes sans soudure destinés principalement au marché européen des équipements mécaniques sont laminés par un producteur ukrainien à des prix compétitifs. » Quelle est donc la stratégie du groupe pour la production nationale ? Je pense à tous ces salariés qui fabriquaient des tubes tubes sans soudure en France et qui sont dans une incertitude insoutenable sur leur avenir depuis des années. Dans une entreprise transparente, qui affiche sa confiance en l'avenir et dont l'État est le principal actionnaire, la stratégie est-elle de laisser au bord du chemin ses collaborateurs de la première heure ?

son marché en matière de fourniture d'équipements pétroliers, pour des raisons que tout le monde comprend. Les différentes entreprises qui ont été confrontées à un tel effondrement de leur marché ont dû prendre des mesures dont vous avez raison de souligner qu'elles ont difficiles. Elles ont mis en évidence un problème de compétitivité de la plateforme France. C'est un sujet sur lequel nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention de la Haute Assemblée et de l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître que,

compétitivité. C'est pour cela que la numérisation des entreprises, c'est-à-dire le fait de transformer leur manière de produire, en augmentant le poids des robots ou des machines à commande additive, est

Aujourd'hui, il en reste 8. La perte progressive des capacités de production sidérurgique ou le rachat des entreprises historiques françaises par des conglomérats, voire des concurrents étrangers, le transfert des talents, des technologies à l'étranger, qui sont tendance alarmante, se retrouvent dans la plupart des pans de notre industrie. Madame la secrétaire d'État, ne croyez pas que nous soyons fatalistes. L'industrie française possède des atouts considérables. Il faut simplement que vous la défendiez sans naïveté face à notre affaiblissement industriel, pour ne pas dire face aux attaques contre notre souveraineté dans certains domaines particulièrement stratégiques. Pourquoi une telle apathie lorsque General Electric, après avoir racheté plusieurs branches d'Alstom, ignore totalement les engagements pris auprès de l'État et annonce de surcroît près de 1 000 suppressions d'emploi ? Je m'interroge lorsque la sucrerie Saint-Louis Sucre, rachetée par des Allemands, s'apprête à cesser la production en Normandie, fragilisant tout l'écosystème local.

économique et social, le FDES. Quand assumerez-vous de vous saisir de tels outils pour soutenir et protéger nos industries stratégiques, clés de notre souveraineté économiques ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Ce combat pour l'industrie, nous le menons, me semble-t-il, sans naïveté. Vous avez cité les investissements étrangers en France et le contrôle que nous opérons : je puis vous assurer, pour avoir un droit de regard sur de telles décisions, que nous bloquons certains actionnaires.

Les fermetures successives de sites et les destructions massives d'emplois sont presque une fatalité. De ce point de vue, les travaux de notre mission d'information ont permis d'apporter un autre éclairage, d'abord en rappelant que l'acier est essentiel à notre économie, en particulier à des filières comme celles du bâtiment, des transports ou même des énergies renouvelables, ensuite en cherchant à analyser les grandes mutations en cours pour mieux préparer l'avenir, plutôt que de revenir sur les erreurs du passé. Afin de construire un avenir durable pour le secteur sidérurgique, je retiendrai qu'un engagement fort de l'État sera nécessaire pour soutenir ce dernier et pallier les défaillances du marché, à travers une politique industrielle à la hauteur des enjeux. Cet engagement de l'État doit avant tout permettre à notre filière sidérurgique de s'inscrire résolument dans la transition énergétique. Avec 19 millions de tonnes de carbone produites chaque année, la sidérurgie représente 4 % des émissions de carbone nationales. Aussi, l'un des grands défis qu'il faudra relever est celui de la décarbonation. Pour cela, il faudra « mettre le paquet » sur la recherche, mais aussi être vigilant sur les fuites de technologie. Ainsi, nous proposons qu'une recherche financée sur fonds publics soit exploitée sur le territoire européen pendant au moins cinq ans. Nous formulons également plusieurs propositions, afin de développer le recyclage et l'écoconception. Outre la contribution au nécessaire développement de l'économie circulaire, le recyclage de l'acier répond à plusieurs impératifs. En l'absence d'une vraie stratégie d'approvisionnement durable et responsable, notre production d'acier reste dépendante de matières premières non disponibles sur notre territoire national. elles pose de lourds problèmes environnementaux, voire éthiques : je pense notamment au cobalt. Enfin, nous nous devons d'anticiper la croissance des besoins dans le secteur des énergies renouvelables. Lorsque nous avons auditionné le directeur de Siemens Gamesa, je lui ai demandé s'il achetait en France l'acier utilisé pour la fabrication d'éoliennes. Il m'a répondu qu'il faudrait pour cela

Valérie Létard, de l'excellente qualité de leurs travaux. Moi-même élue d'un département lorrain, le sujet de la sidérurgie ne peut me laisser insensible. Dans un contexte mondial fortement concurrentiel, la filière sidérurgique doit bien sûr s'adapter. Le verdissement de la stratégie industrielle comme la modernisation des process de production sont de véritables leviers de sa transformation. Je citerai ainsi deux réussites symboliques dans ma région : le projet de transition énergétique de Novacarb, en Meurthe-et-Moselle, et la transformation industrielle du site de Florange.

un mondial de son secteur, elle souffre comme beaucoup de la concurrence asiatique à bas coûts, du protectionnisme américain et de la surproduction mondiale. Dans ce contexte, elle continue toutefois à se moderniser et à innover. Elle a engagé un plan de redressement et d'investissement de 130 millions d'euros qui commence à porter ses fruits, et elle réfléchit aujourd'hui à un partenariat « au partenariat « au nom de la pérennité de l'entreprise et de l'emploi ». Cependant, on ne peut pas dissocier la stratégie industrielle de l'entreprise des leviers à disposition des pouvoirs publics permettant de créer un environnement favorable. Je fais référence ici à l'évolution récente, mais insuffisamment connue, du code des marchés publics, qui permet d'introduire des critères fondés sur l'origine géographique des produits favorisant ainsi le, mais aussi mais aussi à l'introduction de quotas de CO2 dans les règles européennes, ou encore à la taxation des imports extra-européens, un sujet qui revient régulièrement, comme vous le savez. Madame la secrétaire Madame la secrétaire d'État, quelle est la position du Gouvernement sur les quotas de CO2 et sur la taxation des imports de produits hors Union européenne ? Que proposez-vous pour informer et, surtout, rassurer les collectivités, afin qu'elles s'approprient les nouvelles dispositions du code des marchés publics que je viens de mentionner ? La parole est à Mme la secrétaire

ou d'autres éléments qualifiant l'incidence environnementale de la marchandise que vous souhaitez acheter, vous réintroduisez dans l'équilibre de l'offre et dans son appréciation un outil

je vais à mon tour évoquer Ascoval, emblématique dans l'histoire de notre industrie sidérurgique, et ce à double titre. Cette entreprise a été l'un de nos fleurons industriels,

Elle est la preuve qu'il est indispensable que les pouvoirs publics s'impliquent dans la vie économique et fassent preuve de volontarisme pour protéger notre industrie. En effet, Ascoval a été sauvée grâce à l'importance des investissements réalisés- l'État et les collectivités locales lui ont ensemble apporté près de 35 millions d'euros, un soutien financier sans lequel il n'aurait pas été possible de maintenir l'activité du site. Sur ce sujet, le rapport préconise, entre autres, la reconstitution d'un véritable ministère de l'industrie capable de mettre en oeuvre, à travers Bpifrance, des investissements importants. de la récente présentation de son Pacte productif, M. le ministre Bruno Le Maire a surtout évoqué une baisse d'impôts pour les entreprises, mais très peu la question des investissements.

Peut-être est-ce en réponse à cette préconisation que le ministre a récemment évoqué la possibilité de créer un conseil État-régions pour partager les orientations des politiques industrielles nationales et régionales ? Pourriez-vous nous en dire

la France est confrontée à un double enjeu en matière de sidérurgie : la lutte conte le décrochage industriel et la préservation de la souveraineté nationale. D'une part, les emplois de la filière sidérurgique sont menacés ; d'autre part, la souveraineté industrielle est remise en question de manière générale en France.

français. En 1954, les quatre plus grandes sociétés sidérurgiques françaises représentaient environ 50 % de la production nationale. En 2019, près des deux tiers de l'acier produit sur le sol français est issu des usines du seul groupe ArcelorMittal. De fait, plus qu'un marché français, il apparaît évident que la filière sidérurgique en France fait partie d'un marché plus extensif et que, comme le souligne le président de l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, président d'ArcelorMittal France, nous sommes dans un marché européen, l'Europe jouant elle-même dans un marché mondial.

Il reste actuellement 8 hauts-fourneaux actifs en France, alors que l'on en comptait 152 en 1954. Comme le rappelle le rapport, les conséquences sociales et économiques de ce déclin ont été pesantes pour les principaux bassins sidérurgiques français, à savoir le Grand Est et les Hauts-de-France. Ainsi, le nombre d'emplois dans la filière sidérurgique, qui s'est réduit de 20 % au cours des dix dernières années, continue à baisser, tandis que la reconversion des bassins pose de nombreux défis aux acteurs locaux. On remarque effectivement le besoin français et européen d'avoir une filière sidérurgique, notamment en termes d'emplois et de souveraineté.

elles ont un intérêt à viser les segments à plus haute valeur ajoutée, où elles peuvent retrouver de la compétitivité. C'est le mouvement naturel qu'elles essayent d'opérer

pas d'aujourd'hui. Nous ne le répéterons jamais assez : malgré l'actualité et le traitement médiatique réservé à l'industrie de manière générale et à celle de l'acier en particulier, il y a une industrie de l'acier en France Plus de 40 000 personnes travaillent dans ces entreprises, qui produisent notamment des aciers de qualité à haute valeur ajoutée. Ces salariés sont des spécialistes qui font appel à des technologies de pointe.

ni même de Florange, où près de 3 000 personnes n'ont jamais « rien lâché », pour reprendre les mots de mon ami Édouard Martin, et ont continué à être fières des métiers qu'elles exercent. Cela étant dit, je souhaite revenir sur l'un des défis majeurs relevés par le présent rapport l'adaptation nécessaire des producteurs d'acier aux exigences de la transition environnementale. La part de la sidérurgie dans les émissions de CO2 s'élève à 6 % aujourd'hui. À ce stade, les nouveaux procédés de production sur lesquels travaillent les chercheurs mettront, à la condition que les niveaux d'investissement restent élevés, quinze à vingt-cinq ans avant d'être opérationnels. Néanmoins, d'autres projets se déroulent parallèlement comme les projets de capture et de stockage du carbone ou les projets de capture et d'utilisation du carbone. Madame la secrétaire d'État, quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour accompagner et soutenir encore plus fortement la plateforme MetaFensch à Uckange, le projet Valorco, ou encore les projets 3D et Icare à Dunkerque ? L'aboutissement de ces projets est intrinsèquement lié à la sauvegarde et au développement du secteur dans notre pays. La parole

Avec l'évolution du système européen d'émission des quotas pour la période 2021-2030, une augmentation mécanique de la tonne de CO2est à prévoir.

secrétaire d'État, ma question est simple : quelle politique de l'énergie la France veut-elle promouvoir en Europe pour concilier maîtrise des coûts de l'énergie et faibles émissions ? Je connais une énergie qui répond à l'ensemble de ces caractéristiques : c'est l'énergie nucléaire. Quelle est donc la réponse du Gouvernement au rapport remis cette semaine

des processus industriels est une des chaînes de valeur stratégique que nous avons relevée à l'échelle européenne, et qui a été validée comme telle. Elle pourra faire l'objet-

rappelé, nous venons de recevoir le rapport de Jean-Martin Folz qui porte essentiellement sur la situation de l'EPR de Flamanville. Il relève un certain nombre de dérives dérives que nous allons étudier de manière plus approfondie. Le Premier ministre a été assez clair sur le sujet : la question du futur programme nucléaire, s'il y en a un, sera tranchée dans les prochains mois.

En effet, comme dans tout secteur économique, pour rester compétitives, voire développer leurs activités, les entreprises de la filière sidérurgique ont besoin de lisibilité quant à leurs dépenses. En premier lieu, il y a la dépense imposée, notamment la compensation qui leur est demandée pour leurs émissions de CO2, compensation qui est à présent inéluctable pour une évolution rapide vers les adaptations technologiques permettant de réduire ces émissions à leur minimum. Il est nécessaire et urgent que ces entreprises puissent avoir une visibilité suffisante Pour cela, une feuille de route claire doit leur être donnée concernant les quotas et le prix à la tonne avec un horizon à cinq ans, afin de leur permettre d'anticiper ces importants surcoûts de production. Qu'est-il prévu par le Gouvernement à ce sujet ? Par ailleurs, pouvez-vous nous faire un point précis sur la mise en place aux frontières de l'Europe d'un possible test sur la filière acier du mécanisme d'inclusion carbone en remplacement du système actuel des quotas ETS ? En second lieu, la visibilité sur le coût de l'énergie, et plus particulièrement de l'énergie électrique, est primordiale sur un marché qui fluctue beaucoup et sur lequel les mécanismes d'économies

Pour terminer, je me permettrai une remarque : diminuer l'empreinte carbone de la sidérurgie suppose aussi de s'attaquer aux transports des matières premières et des produits finis. Or, vous le savez, le multimodal est très difficile à mettre en oeuvre, la SNCF restant très frileuse sur ce sujet. Aussi, la filière est prête à s'organiser en ce sens, mais elle attend des dispositifs d'aide lui permettant de développer cette intermodalité et de diminuer ainsi les émissions carbonées des camions. Madame la secrétaire d'État, quelle est votre vision à ce sujet ?

sur deux jambes. Le numérique, la nouvelle économie, l'intelligence artificielle, la robotisation, oui ! Mais notre industrie doit leur emboîter le pas. Vous en êtes convaincue, donc que l'on vous en donne les moyens, que l'on dise enfin que l'industrie est une priorité nationale. Combien de territoires s'interrogent sur le devenir de leurs entreprises industrielles ? On a parlé

ministre de l'industrie doit avoir les moyens d'être l'interlocuteur privilégié, identifié, pour faciliter la tâche des acteurs industriels et transformer le contenu des contrats stratégiques de filière. En effet, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. Les moyens doivent être

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 18 octobre 2006, Françoise Férat présentait à notre commission de la culture, dont elle était alors membre, un rapport sur la place de l'enseignement agricole dans le système éducatif français. Il plaît au Sénat de prendre appui sur ces travaux de fond pour évaluer régulièrement l'état et les évolutions des politiques publiques. Le présent débat n'a d'autre ambition que de poser les termes généraux d'un bilan, qui devra nécessairement être prolongé. La question posée est très générale pour permettre aux sénatrices et aux sénateurs qui nous font l'honneur de leur participation de s'exprimer librement sur des sujets d'ampleur ou des situations locales. Depuis 2006, le système éducatif français n'a cessé d'évoluer et de se transformer. Les révisions ont succédé aux réorganisations administratives, et les plans d'économies aux mesures d'optimisation ou de rationalisation, qui ont souvent affaibli un réseau d'établissements toujours aussi fragiles. Les deux années qui viennent de s'écouler n'ont pas été épargnées par le maelström de la réforme permanente. Les nouvelles dispositions relatives à l'accès à l'enseignement supérieur contenues dans la loi Orientation et réussite des étudiants, les changements majeurs imposés à l'ordonnancement du baccalauréat, des études dans le cadre du lycée et de l'apprentissage ont eu des conséquences très importantes sur l'enseignement agricole. nous ne pensons pas que ses spécificités aient été pleinement considérées et préservées. Le sentiment qui prédomine est, au contraire, celui d'un nouvel affaiblissement de ses capacités, de ses moyens et de sa notoriété. Dans le très vaste ensemble du service public de l'éducation, il nous semble que l'enseignement agricole demeure la cinquième roue du tracteur. En 2006, notre collègue Françoise Férat considérait qu'il était à la croisée des chemins ; après toutes ces réformes, on peut se demander s'il n'est pas dans l'ornière L'ambition de ce débat est d'apporter une première contribution à un inventaire nécessaire. Avant d'aborder nos divergences, soulignons nos consensus. en tant qu'historien de l'agriculture, que la ruralité n'est pas ce monde immobile, bloqué par la routine et incapable de participer activement aux évolutions de la société parfois décrit par ceux qui le regardent avec dédain et condescendance. Ce mépris participe d'une incompréhension croissante entre les villes et les campagnes et, au sein de ces dernières, entre ceux qui y vivent et ceux qui les cultivent. Notre pays, par ses traditions et par l'importance de sa ruralité, ne peut accepter que ce dissentiment persiste et s'aggrave. L'enseignement agricole est un des moyens de réparer ce lien qui menace de se rompre. Depuis la révolution néolithique, les agriculteurs- les paysans, comme j'aime à les appeler -ont su adapter en permanence leurs productions, leurs pratiques et leurs organisations sociales aux évolutions de la consommation, des goûts et des habitudes alimentaires, de même qu'aux changements climatiques et aux bouleversements géopolitiques. Reste que jamais dans cette longue histoire les mutations de l'agriculture n'ont été aussi profondes,

mais une autre la remplace, qui devra trouver les ressources nécessaires pour affronter des enjeux majeurs. Le premier de ces enjeux est climatique. Le deuxième, social, car il faut trouver les moyens de faire vivre ensemble, dans l'espace rural, des populations qui n'ont pas la même utilisation des sols des sols et des ressources naturelles. Les enjeux sont aussi évidemment environnementaux et économiques. Dans cet hémicycle, nous partageons une même conviction : l'enseignement, la formation et la recherche seront déterminants pour accompagner, guider et éclairer ces mutations majeures. Le renforcement et le développement de l'enseignement agricole à tous ses degrés doivent donc devenir une cause commune et une obligation de l'État ! Au reste, l'affirmation de cette nécessité n'est pas nouvelle.

avancées ont été oubliées, et l'Observatoire national de l'enseignement agricole a été remplacé par l'Observatoire de l'enseignement technique agricole, aux compétences réduites et qui ne rend plus de rapport Parmi ses recommandations, l'Observatoire national de l'enseignement agricole avait insisté sur l'importance des dynamiques de déconcentration et de décentralisation pour favoriser les relations entre les services déconcentrés du ministère de l'agriculture, les rectorats, les conseils régionaux et tous les professionnels.

doivent maintenant se financer par le biais des contrats qui leur sont proposés. La capacité des collectivités territoriales à aider, par la formation, des filières agricoles à subsister ou à se construire en a été considérablement réduite. Il nous faut évaluer les conséquences de cette dépossession. autre motif d'inquiétude concerne les exploitations agricoles gérées par les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Leur situation économique s'est dramatiquement dégradée, et la moitié d'entre elles seraient aujourd'hui en quasi-faillite. Je rappelle que la loi donne à ces établissements trois missions essentielles et indissociables : assurer la formation par la pratique, participer à l'animation et au développement des territoires et contribuer aux activités d'expérimentation et de recherche appliquée. L'enseignement agricole a la difficile mission d'éveiller l'intelligence de la main et de l'outil et de donner les bases d'une compréhension globale et souvent empirique de systèmes rendus complexes par les interactions fortes entre le végétal, l'animal, la nature et l'humain en société. Ces savoirs ne sont malheureusement pas les plus valorisés par notre système éducatif. Permettre aux établissements d'enseignement agricole d'en assurer la promotion et la transmission dans les meilleures conditions est donc un enjeu majeur pour lequel l'engagement de l'État doit être sans faille,

-ont joué un rôle essentiel comme structures de soutien aux agriculteurs, aux filières professionnelles et,, aux territoires ruraux. J'évoquerai l'histoire de l'école d'agriculture et des industries rurales de Neuvic, en Corrèze, qui permettait aux élèves, après leur scolarité, de mener une partie de leur activité au sein d'une structure associée à l'école et gérée comme une coopérative. Un lien fort était ainsi tissé entre l'école, les professionnels et les terroirs. Il faut aujourd'hui préserver et développer cette interaction fondamentale, car c'est un levier efficace d'aide à l'agriculture dans sa nécessaire mutation. Pour que cette politique soit active, il faut que l'enseignement agricole reste attractif. Or, je le répète, il n'est pas du tout assuré que les réformes du baccalauréat et de l'accès à l'enseignement supérieur aient renforcé Les rares statistiques disponibles semblent montrer au contraire qu'il a eu à pâtir d'une concurrence accrue avec les filières générales. Avec la nouvelle organisation des études de la classe de terminale, l'enseignement de l'agronomie est assuré dans le cadre d'une option, non d'une spécialité. Les heures de cours consacrées à cette matière vont donc globalement diminuer, et il est à craindre que les élèves qui souhaitent prolonger leur cursus dans le supérieur ne se détournent de l'enseignement agricole au profit d'autres lycées, d'autant que très peu de lycées agricoles ont retenu cette option. Mon inquiétude majeure concerne les bacheliers des filières technologiques et professionnelles. Comme l'a dénoncé le Défenseur des droits, ces élèves ont été massivement écartés de l'enseignement supérieur par la procédure Parcoursup. Nous avons absolument besoin de savoir ce que sont devenus ces bacheliers issus de l'enseignement agricole. Pour demeurer attractif, il faut que cet enseignement offre la possibilité d'une poursuite d'études au-delà du baccalauréat.

personnels ont aujourd'hui besoin d'une reconnaissance à la mesure de leur engagement exceptionnel. Ils sont trop nombreux à travailler dans la précarité et à être bloqués dans leur carrière par des statuts d'emploi qui leur interdisent toute mutation.

Alors même que, après plusieurs années de recul des effectifs, le nombre d'élèves va augmenter, cette hausse, souhaitable pour le monde agricole et, plus largement, pour l'ensemble de notre société, va donc être accueillie par une dégradation de la qualité de l'accueil, avec d'inévitables conséquences sur celle de l'enseignement. Le relèvement des seuils de dédoublement est particulièrement néfaste à nos yeux. Ainsi, comment imaginer réaliser des travaux pratiques dans de bonnes conditions avec des effectifs augmentés d'au moins trois élèves, quand il s'agit, par exemple, de manier des outils dangereux,

; on peut facilement imaginer ce qu'il en adviendra sous la pression de restrictions budgétaires malheureusement constantes ... Avec, à la clé, des problèmes extrêmement concrets, comme celui des salles informatiques

à faire choisir aux élèves deux enseignements de spécialité et deux enseignements optionnels spécifiques à l'agriculture, certaines disciplines fondamentales étant d'ailleurs dispensées sous forme optionnelle. Dans les faits, les diminutions de moyens, en termes tant de dotation horaire globale que de postes, conduisent à choisir entre enseignements de spécialités et options facultatives. Celles-ci permettent pourtant aux jeunes

une large intersyndicale a eu beau interroger vos services à de nombreuses reprises sur cette question, rien n'y a fait ! J'aimerais évoquer maintenant, trop brièvement, les lycées professionnels maritimes, qui témoignent de la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. Critique, car le métier de marin-pêcheur connaît lui aussi une crise de recrutement, en partie liée à un manque de considération pour ces formations. Ainsi, depuis 2007, les effectifs de marins-pêcheurs ont chuté de 14 %. Même dans les familles de ces professionnels, on observe un assèchement des recrutements. En cause, comme le fait apparaître le récent rapport de notre collègue député Sébastien Jumel, la mauvaise image de la voie professionnelle, mais aussi un maillage territorial insuffisant, avec seulement douze lycées professionnels maritimes, et surtout des moyens qui ne permettent pas d'accueillir les lycéens en pension complète. Cela conduit ces établissements à recruter quasi exclusivement des jeunes présents sur leur territoire, quand beaucoup d'autres, en recherche de formation, mais éloignés, pourraient s'y épanouir. Il en va de même pour le contenu des formations dans le cas de la voie professionnelle. Par exemple, les exigences de la pêche durable ne sont enseignées que sous la forme de réglementations à respecter ou d'une courte sensibilisation en classe de seconde, alors que cette dimension devrait faire partie intégrante de la formation, avec des sorties sur le terrain et des rencontres avec l'Observatoire de la biodiversité marine, comme dans le cadre du BTS Pêche et gestion de l'environnement marin. Telle est, hélas, l'ambition du Gouvernement pour l'enseignement agricole, à plus forte raison lorsqu'il est professionnel, pour les territoires ruraux où il se situe bien souvent et pour des métiers pour la plupart en souffrance. L'exemple de la pêche, sur lequel je me suis attardée, car il est trop rarement évoqué, permet de prendre conscience de ce qui se joue.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1850, à Nancy, une statue fut érigée à la mémoire de Mathieu de Dombasle, et la place sur laquelle elle se trouve porte désormais le nom de ce Lorrain considéré comme le père de l'enseignement agricole. agricole. Animé par l'envie de transmettre sa passion, cet agronome avait bien compris que l'enseignement agricole ne visait pas seulement à améliorer les techniques et à augmenter la productivité il avait compris que le travail de la terre donne à l'homme une activité noble, par laquelle tout un chacun peut s'élever. C'est dans cet esprit que l'enseignement agricole s'est développé en France pendant plus de deux siècles. Cet enseignement connaît aujourd'hui des formes diverses, du secteur public au secteur privé en passant par les maisons familiales rurales et l'apprentissage en alternance. Ces formes constituent un ensemble riche et complémentaire, dont la diversité fonde l'excellence de la filière.

La loi attribue à cet enseignement différentes missions, qui vont bien au-delà de la seule formation scolaire et professionnelle. Il doit également contribuer à l'animation du territoire, à la coopération internationale, à l'expérimentation et à l'insertion. C'est dire l'importance que la puissance publique lui confère et surtout la responsabilité qui incombe aux acteurs de terrain qui le font vivre au quotidien dans nos territoires. La France, en tant que première agriculture européenne, doit savoir évoluer pour conserver sa place sur les marchés internationaux, alors que d'autres modes de consommation et d'autres types de besoins émergent. L'évolution de l'agriculture face à celle du climat, aux impasses techniques et technologiques et aux limites de l'efficacité de la chimie, et avec le développement du bio, de l'agroécologie et des marchés de proximité, oblige tous les acteurs agricoles à adapter leurs savoirs

imposent de nouvelles exigences en matière d'innovations techniques et d'adaptation technologique, donc aussi en matière pédagogique. Nouveaux besoins, nouveaux publics, nouveaux savoirs : l'enseignement professionnel agricole, à l'image du secteur, à l'image du secteur, devra nécessairement évoluer pour perdurer et maintenir son attractivité et son excellence. Si une grande partie du travail échoit directement aux professionnels, les pouvoirs publics ont évidemment un rôle important à jouer.

Cette agilité est une spécificité importante de l'enseignement agricole. Ensuite, il importe de renforcer les moyens consacrés à l'enseignement agricole.

des générations, enjeu essentiel, car un agriculteur sur deux a plus de 55 ans. L'accueil du public hors cadre familial est donc indispensable pour assurer l'avenir de notre agriculture. chers collègues, investir dans l'enseignement professionnel agricole, c'est investir tout à la fois dans notre souveraineté alimentaire, dans la transition écologique et dans la cohésion de nos territoires. Au début du XXI siècle, alors que l'humanité fait face à de nouveaux défis, il est essentiel de nous souvenir du message de Mathieu de Dombasle : l'enseignement agricole est avant tout un enjeu de transmission, dans lequel l'humain joue un rôle central. Dans cette perspective, l'enseignement professionnel agricole doit contribuer à ce que notre société renoue un lien apaisé avec son agriculture, qui en a bien besoin ! La parole est à Mme Dominique Vérien.

permettant à des élèves qui ne se sentent pas à leur place dans l'enseignement général ou dans l'éducation nationale de se retrouver pour ainsi dire en famille, encadrés, guidés, accompagnés vers la réussite. Malheureusement, le critère d'âge des stages dans l'enseignement professionnel limite aux enfants de plus de 14 ans l'accès à ces maisons,

Autant de raisons qui rendent cet enseignement indispensable pour la diversité des modes d'enseignement et la réussite du plus grand nombre de nos jeunes. voilà : la réussite de cet enseignement, si elle n'est pas limitée aux secteurs ruraux, y est tout de même concentrée. Or c'est là que le bât risque de blesser dans la filière de l'apprentissage. En effet, les régions contribuaient souvent,

D'autant que ce centre doit affronter une autre difficulté : il ne trouvera bientôt plus d'apprentis dans nos communes, celles-ci devant financer 50 % du coût de la formation depuis le retrait de la compétence La réussite de cet enseignement tient aussi à la qualité des enseignants. Or, notamment dans le secteur privé de l'enseignement agricole, vous vous étiez engagé, monsieur le ministre, à revaloriser la grille indiciaire des enseignants agents de catégorie 3 et à ouvrir plus largement

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'enseignement agricole a une véritable histoire, avec des missions qui lui sont propres. propres. Enseignement général et technique, il comprend à la fois des stages en exploitation et une ouverture socioculturelle. L'enseignement agricole privé occupe une place importante dans le dispositif et l'offre éducative. Quant aux maisons familiales rurales, elles sont une vraie spécificité, avec des formations par alternance. L'enseignement agricole a su montrer ses facultés d'adaptation à l'évolution de l'agriculture, à la modernisation de celle-ci au long du XX siècle. Il a évolué avec la révolution technique et le passage du travail avec cheval et attelage à une mécanisation poussée, parfois exagérée. Or, depuis une vingtaine d'années, un décalage, une fracture sépare l'évolution de la société et l'adaptation de l'enseignement agricole. La société est téléguidée vers une image de l'agriculteur pollueur, voire criminel, l'utilisation des réseaux sociaux comme canal de communication au service d'une définition outrancière du bien-être animal et d'une alimentation bio et durable. Si certains médias mettent l'accent sur les dérives et dénoncent abus, l'agriculteur aime son travail et ses animaux ; il est passionné par son métier. L'agri-bashingdéveloppé par notre société porte aujourd'hui un vrai préjudice à la profession agricole, ainsi stigmatisée. L'enseignement agricole s'en trouve modifié et dogmatisé vers des filières environnementalistes en décalage avec une grande partie de la profession. Or, pour rester attractif, il doit rester ouvert à tous les types d'agriculture. Voilà une trentaine d'années, 90 % des élèves étaient d'origine agricole et rurale et avaient un véritable projet d'installation ; aujourd'hui, ils ne sont plus que 30 % environ dans ce cas. Bien sûr, les autres 70 % sont sensibilisés aux notions agricoles, mais pas au milieu agricole et à son environnement naturel. L'enseignement agricole a formé ces dernières années des jardiniers de la nature qui viennent malheureusement gonfler les chiffres des demandeurs d'emploi ... L'agriculture dite conventionnelle doit reprendre sa place dans le dispositif éducatif, tout en intégrant, bien sûr, les éléments du développement durable. l'enseignement agricole retrouvera ses lettres de noblesse en conduisant à l'installation de jeunes agriculteurs pour toutes les agricultures, en formant de jeunes agriculteurs qui soient de véritables chefs d'exploitation, des chefs d'entreprise compétents en gestion et en technologie. les établissements agricoles, lycées professionnels publics ou privés et maisons familiales rurales, sont de véritables outils d'aménagement du territoire. Leurs objectifs pédagogiques sont centrés sur les productions et spécificités régionales. régionales. Je pense aux filières viticoles dans le Bordelais et en Alsace et aux filières laitières, fromagères et productions animales dans le Massif central et les Alpes. Ce potentiel de richesse pédagogique régionale et locale doit être renforcé, valorisé et ainsi offrir une véritable plus-value à l'enseignement agricole.

! Cessons donc cet agri-bashing destructeur, qui a de fortes conséquences sur l'avenir de l'enseignement agricole et la formation des jeunes ! L'enseignement agricole a toujours été à la pointe en matière d'évaluation des jeunes

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quel avenir pour l'enseignement agricole ? Il s'agit là d'un sujet important, comme les précédents orateurs l'ont souligné, pour les territoires ruraux, mais aussi pour l'ensemble du pays, au regard des enjeux auxquels nous sommes confrontés sommes confrontés comme des perspectives que nous offre l''agriculture urbaine. Nous parlons de 200 000 élèves à la rentrée scolaire dernière, accueillis au sein de 800 établissements publics et privés dispensant des formations initiales, des formations permanentes et des formations par alternance.

Quels sont les enjeux de cet enseignement ? S'agissant des métiers liés à l'activité agricole, les formations doivent permettre de favoriser la reprise des exploitations, qui constitue un des enjeux majeurs, en accueillant notamment des néo-agriculteurs.

prendre en considération la multifonctionnalité de l'agriculture en intégrant les enjeux environnementaux dans les pratiques agricoles, notamment la biodiversité, l'eau, les paysages, et de mettre ainsi en oeuvre le nouveau paradigme de l'agroécologie. Il s'agit également de s'adapter aux évolutions climatiques et de saisir les opportunités en matière d'énergies renouvelables à partir de la biomasse. À cela s'ajoute le développement de la numérisation, de l'automatisation, mais également de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour ce qui concerne les métiers des territoires ruraux, de manière plus large, les établissements d'enseignement constituent très clairement des outils de développement local au travers non seulement des compétences qu'ils dispensent, mais aussi de leur capacité à participer à la conception et à la mise en oeuvre des projets territoriaux. Au-delà de l'agriculture, il est donc nécessaire que ces établissements adaptent les formations aux caractéristiques de leur territoire, afin de favoriser la mise en oeuvre de leur potentiel. Ces établissements offrent par ailleurs des formations nécessaires pour répondre aux besoins croissants

rapidement un travail à l'issue des formations qu'il dispense. Quels challenges doit relever l'enseignement agricole pour qu'il tienne les promesses faites ? Il doit continuer à s'adapter aux évolutions des savoirs nécessaires et renforcer ses capacités à expérimenter. Il faut promouvoir les formations proposées et faire connaître les gisements d'emplois importants qui existent dans le domaine agricole et dans les métiers des campagnes. Pour ce faire, l'enseignement agricole doit disposer de moyens budgétaires

De ce fait, aujourd'hui, les établissements sont confrontés à de réelles difficultés financières, alors même que de nombreuses exploitations tenues par ces établissements ont besoin de réorganisation et de recapitalisation. Les dotations globales horaires qui ont diminué qui ont diminué ont été compensées par le relèvement des effets de seuil, ce qui ne peut qu'avoir des effets négatifs sur la qualité de l'enseignement dispensé. Les perspectives ne sont pas encourageantes, puisqu'il semblerait qu'une poursuite de ces réductions de 2 % par an jusqu'en 2022. De plus, la réforme de l'apprentissage, avec une large ouverture au privé, est de nature à renforcer les difficultés financières des établissements publics qui accueillent 75 % des apprentis ; à cet égard, les centres de formation

il s'agit bien là de l'originalité de l'enseignement agricole. En conséquence, il apparaît évident que l'enseignement agricole peut participer fortement au renouveau des campagnes françaises que l'on constate, et dont témoigne la croissance démographique

Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, notre agriculture manque de bras. La situation est tendue : 70 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues, et les agriculteurs font de plus en plus appel à des sociétés qui font travailler de la main-d'oeuvre étrangère. Pourtant,

La réalité est, en fait, tronquée. Depuis plus d'une décennie, la filière des services à la personne a supplanté les filières de production : parfois, certains lycées agricoles n'ont d'agricole que le nom.

Derrière ces changements de formation-vous l'aurez compris-, se cachent des enjeux d'image. Ils reflètent également la mutation de notre ruralité, qui est de moins en moins agricole : les filles et les fils de paysans, ne voulant plus reprendre les exploitations, désertent ces filières-comme cela a été dit, seulement un élève sur dix est un enfant d'agriculteurs. Se poser la question de l'avenir de l'enseignement agricole, c'est donc inévitablement se poser celle de l'avenir de notre agriculture et de son attractivité pour les jeunes. le contexte. Les lycées agricoles, qui se distinguent des autres lycées professionnels sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, ont notamment pour mission de participer à l'animation et au développement des territoires. En 1984, date de la loi Rocard, cet enjeu avait toute sa portée, car les lycées agricoles formaient majoritairement des enfants d'agriculteurs ou des jeunes qui voulaient le devenir. Aujourd'hui, la donne a changé puisqu'ils forment à d'autres métiers que la production agricole. Cela entraîne des conséquences, relevées notamment par le Conseil national de l'enseignement agricole privé. Ses responsables indiquent : « L'avenir de l'enseignement agricole sera pleinement pris en compte par les acteurs locaux quand sera mieux reconnue sa capacité de satisfaire certaines des politiques publiques territoriales. Il s'agit de changer de regard et de considérer désormais les lycées agricoles comme des partenaires des politiques publiques territoriales en leur donnant les moyens de réaliser cette interface entre monde économique, population et éducation des jeunes ou des adultes en formation continue. Ces lycées sont des centres de ressources pour les territoires. » Ceci me semble essentiel : il est primordial de coller aux besoins des territoires, car leurs mutations démographiques, sociologiques, économiques, paysagères et environnementales affectent directement l'avenir de l'enseignement agricole.

Tous présentent des caractéristiques communes : la capacité à l'encadrement d'équipe, car le salariat va se développer, les circuits courts, les métiers de la médiation, le conseil en agroécologie, les compétences en analyse de données, la e-maintenance et la compétence prédictive, les métiers de la qualité Autant d'horizons pour demain. Mais à quoi serviront nos techniciens agricoles, nos ingénieurs agronomes, nos experts en organisation si notre agriculture se meurt ? Quel avenir pour ces diplômés ? On en revient à la question préalable de l'avenir de notre agriculture, car on ne maintiendra pas une agriculture sans agriculteurs.

les aléas climatiques et sanitaires, et des prix d'achat non rémunérateurs. La véritable question est la suivante : comment redonner une image attractive à ce métier ? Que dire aux jeunes pour leur donner l'envie de s'installer ? Comment inciter l'éducation nationale à valoriser cette filière dans ces conditions ?

me l'a confirmé, en indiquant que les filières paysagères ou concernant les soins de chevaux plaisent plus, car le métier visé paraît moins dur et l'image bien meilleure. Quel désastre ! Comment en sommes-nous arrivés à ce point de dénigrement de notre agriculture ?

En effet, au-delà des préoccupations budgétaires, devenues centrales ces dernières années, un climat de malaise s'installe peu à peu chez l'ensemble des acteurs et partenaires de l'enseignement agricole. » Elle y préconisait notamment ne plus tenir l'enseignement agricole à l'écart des procédures d'orientation des élèves et de promouvoir une image plus moderne et attractive des filières et des métiers. Treize ans plus tard, les préconisations pourraient être les mêmes, car si l'enseignement agricole a su adapter

Nous sommes tous coresponsables de cette baisse d'attractivité : agriculteurs, organisations professionnelles, syndicats, éducation nationale. Nous avons tous lâché prise. Et nous nous sommes arrangés pour que l'enseignement agricole survive. L'Occitanie a su renverser cette tendance en menant une politique de cohérence sur l'analyse des formations et de leur implantation, en concertation notamment avec les chambres d'agriculture. Les vraies réponses à la question de l'avenir d'un enseignement redevenu agricole passeront forcément par un travail sur la juste rémunération des agriculteurs, car notre agriculture répond à des enjeux transversaux et fondamentaux pour coller coller à l'attente sociétale : santé publique, environnement, économie, aménagement du territoire, évolution des goûts des consommateurs. Il faut absolument penser notre politique agricole de son enseignement à la production en adoptant une stratégie à la hauteur de ces enjeux,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à quoi ressemblera le lycée agricole de 2040 ? En tant que rapporteur sur les crédits de l'enseignement technique agricole, je remercie mes collègues du CRCE de nous inviter à nous pencher sur cette question. Permettez-moi tout d'abord de porter un regard positif. Fruit d'une longue tradition, l'enseignement agricole n'a plus et ne pourrait plus avoir la même vocation qu'hier : il est devenu un enseignement en prise avec les défis émergents. De l'information donnée au consommateur à la question du glyphosate en passant par celles du bien-être animal, du bio, ou encore de l'épandage des pesticides à proximité des habitations, nous le voyons, l'agriculture et, par extension, l'enseignement agricole se trouvent à la croisée de profondes préoccupations sanitaires et environnementales. enseignement ne regarde pas le train passer. Aujourd'hui, quatre élèves sur dix étudient les services à la personne. Ce fait marquant résume les profonds changements de l'enseignement agricole au cours de ces dernières décennies. telle évolution reflète aussi celle du monde rural, où le poids des agriculteurs recule. Seuls 12 % des élèves sont enfants d'agriculteurs, alors qu'ils constituaient plus de 40 % des effectifs trente ans plus tôt. De même, les élèves sont de plus en plus jeunes, et la parité est désormais engagée. À cet égard, le budget pour 2020 intègre pour la première année un indicateur d'égalité femmes-hommes qu'il convient de saluer. Il s'engage également dans l'école inclusive. Enfin-c'est là une évolution essentielle-, la passerelle vers l'enseignement supérieur est de plus en plus empruntée : plus de 30 % des diplômés d'un bac pro poursuivent désormais leurs études en BTSA, L'enseignement agricole jouit aussi d'un taux d'insertion professionnelle nettement plus élevé que la moyenne nationale. Si l'on y ajoute le taux de réussite aux examens passant la barre des 85 %, cette filière apparaît comme un choix séduisant pour les élèves. Mes remarques porteront sur des pistes pour améliorer la situation. Nous le savons, les effectifs ne sont pas à la hauteur des espérances, et l'enseignement agricole reste miné par un réel manque d'attractivité. À chaque examen budgétaire, je rappelle dans cet hémicycle l'impérieuse nécessité de rompre avec l'idée répandue selon laquelle l'enseignement agricole serait une voie de garage réservée aux jeunes en situation d'échec. Il est sans nul doute une école de la deuxième chance incroyable, mais il est aussi et surtout une filière d'excellence. Les raisons de ce manque d'attractivité sont connues l'implantation traditionnelle de l'enseignement agricole dans des régions enregistrant une baisse démographique, et, la sous-représentation où la demande existe ; et surtout, le défaut de notoriété auprès de nos jeunes. Combien de collégiens savent que l'on peut devenir ingénieur en intégrant une classe de première technologique agricole ? Combien savent qu'un élève de terminale professionnelle agricole a 59 % de chances de trouver un emploi, contre 42 % pour son homologue de l'enseignement Pour répondre à cette problématique, vous avez lancé, monsieur le ministre, la campagne de promotion L'Aventure du vivant à l'occasion du dernier salon de l'agriculture. Peut-être pourrez-vous nous dire quelques mots sur les résultats attendus de cette campagne, ainsi que sur la manière de mieux communiquer sur la diversité des métiers auxquels prépare l'enseignement agricole. On ne le dit pas suffisamment : l'enseignement agricole permet d'accéder à plus de 200 métiers dans le domaine de l'agriculture et de la nature, et à 280 exploitations et ateliers sur tout le territoire.

c'est le cas dans le secteur de l'agroéquipement. Par ailleurs, l'enseignement agricole est pleinement engagé dans la mise en oeuvre des réformes des baccalauréats général et technologique, de la voie professionnelle et de l'apprentissage. Les établissements pourront désormais élaborer l'offre de formation la plus adaptée aux spécificités locales. C'est le point essentiel sur lequel je vais insister. Cet enseignement doit jouer un rôle prépondérant dans la valorisation de nos territoires en s'articulant autour de projets locaux-je pense bien évidemment aux zones rurales, mais pas seulement. Il constitue aussi un levier incontournable pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire des territoires d'outre-mer, tournés depuis trop longtemps vers l'importation. À cet égard, l'accord conclu en 2018 avec les familles de l'enseignement privé en termes de financement est fondamental. Accueillant environ 60 % des élèves, les établissements privés sont une composante majeure de l'enseignement agricole, au rayonnement et au dynamisme duquel ils contribuent. Il s'agit également de leur donner les moyens de leur développement, alors qu'il existe dans de nombreux territoires d'importants besoins. Signe que l'enseignement agricole tend à s'adapter aux enjeux de notre société, l'année 2020 sera marquée par la mise en oeuvre du plan Enseigner à produire autrement, axé pour l'essentiel sur les transitions et l'agroécologie. Cependant, être en prise avec des défis d'aujourd'hui, c'est également mieux armer les futurs agriculteurs. Par-delà les attentes des consommateurs, l'acte de production devient lui aussi de plus en plus complexe en raison des réglementations changeantes, des pratiques techniques pointues et des incertitudes économiques. C'est pourquoi l'enseignement agricole doit mieux préparer ceux qui se destinent à la gestion d'une exploitation. La volatilité des prix, la gestion des risques, ou encore l'agriculture numérique sont autant de sujets auxquels nous devons sensibiliser les étudiants. les étudiants. Je m'interroge, monsieur le ministre, sur l'installation des jeunes agriculteurs : les établissements ne doivent-ils pas prendre toute leur part dans ce processus ? Je pense en particulier aux territoires ultramarins où, nous le savons, la question foncière est un noeud gordien. Monsieur le ministre, l'enseignement agricole doit sortir d'une logique de conservation et de repli pour entrer dans une logique d'expansion. Alors que nous nous interrogeons sur son avenir, je crois qu'il nous faut prendre conscience que la manière dont nous nous investirons dans ce domaine

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, traiter de l'enseignement agricole, c'est avant tout s'enquérir de l'agriculture de demain. Avec près de 75 % des apprentis dans 806 établissements scolaires, l'enseignement agricole public et privé, filière d'excellence, tient une place essentielle dans le développement de l'apprentissage. Or les récentes réformes de l'apprentissage et du baccalauréat sont porteuses de profondes mutations pour ce secteur. La réforme de l'apprentissage, visée par la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, prévoit ainsi un véritable choc

salariés préparant à un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac verront leurs aides rassemblées et revalorisées, l'aide pour les diplômes supérieurs a pour sa part été supprimée. Or aujourd'hui le diplôme le plus recherché de la filière agricole est le BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, dans la mesure où il permet l'embauche de salariés hautement qualifiés et offre des perspectives de reprise d'installation à terme. Dès lors, la suppression des aides fléchées pour les TPE vers les diplômes post-bac risque de pénaliser une profession qui cherche pourtant à monter en compétence. Un autre questionnement voit également le jour à la faveur de cette réforme : le développement, certes souhaité, de l'apprentissage conduira les lycées à développer des classes mixtes mêlant apprentis et élèves en voie scolaire. Si aujourd'hui les enseignants sont ouverts à cette éventualité en dépit de contraintes pédagogiques supplémentaires, de nouvelles difficultés pourraient apparaître dans la mesure où les enseignants ne sont pas habilités statutairement à intervenir auprès d'apprentis. Il est donc à craindre que dans un avenir proche cette situation ne soulève de nouveaux obstacles qui n'ont pour l'heure pas été pris Enfin, je souhaite évoquer la question de la réforme du baccalauréat général. Cette réforme a permis, je le rappelle, de regrouper les filières S, ES et L. Ainsi, les élèves issus de filières générales pourront désormais choisir parmi douze enseignements proposés, trois spécialités en première, puis deux en terminale.

Cette restriction risque encore une fois d'accroître la déperdition d'élèves s'orientant vers les filières agricoles et, à terme, de mettre en danger l'existence même de celles-ci. En effet, de nombreux jeunes, incertains quant à leur orientation- ils représentent 50 % des élèves détenteurs d'un baccalauréat-, préféreront s'orienter vers des filières proposant un plus large choix d'enseignement. Sans pour autant réclamer le même nombre de choix de disciplines, les lycées agricoles souhaiteraient donner la possibilité à leurs étudiants de suivre des enseignements tels que les sciences économiques et sociales, ou encore le numérique et les sciences informatiques, qui s'inscrivent en totale cohérence avec la révolution technologique du monde agricole et des métiers de l'agriculture de demain.

Au vu de toutes ces interrogations, pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, si votre gouvernement a pris en considération ces problématiques, et, le cas échéant, si des ajustements sont prévus ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, et celle d'aujourd'hui ne sera sans doute pas celle de demain. Quelle agriculture voulons-nous ? Quel rapport à l'environnement, à la consommation voulons-nous ? Pour répondre à ces questions, l'enseignement agricole jouera un rôle décisif. Les défis sont nombreux : comment mieux appréhender les aléas climatiques, les crises sanitaires ? Il est important que l'ensemble de nos exploitations puisse tirer bénéfice de nouvelles technologies, notamment avec l'utilisation des datas, des drones, ou encore de la méthanisation. Pour produire différemment, il faudra être capable d'enseigner différemment. est vrai, monsieur le ministre, que cela a un coût qu'il faut être capable d'assumer dès maintenant. L'enseignement agricole a longtemps fait preuve d'une forte capacité d'adaptation, avec des offres de formation de plus en plus variées. Néanmoins, aujourd'hui, il est important de mieux structurer et de mieux articuler ces offres, notamment en renforçant les passerelles avec l'enseignement dit général. Cela est d'autant plus important que les reconversions professionnelles Cette multitude d'offres nous oblige à une plus grande visibilité sur les différents parcours et leurs débouchés. L'enseignement agricole va du CAP à la licence. Il concerne bien sûr les céréaliers et les éleveurs, mais pas seulement.

Cependant, encore faut-il connaître ce site ... Une meilleure communication est par conséquent nécessaire, afin que ces formations soient connues non pas seulement par une poignée d'initiés, souvent d'ailleurs eux-mêmes issus du milieu agricole, mais bien par l'ensemble de nos étudiants. Près de 80 % des élèves diplômés ne seront pas eux-mêmes agriculteurs à proprement parler. C'est dire à quel point le monde agricole est vaste. Les conseillers d'orientation doivent être mieux informés, tant il existe des formations spécifiques dans chaque région. est important de mener cette démarche, car, avec le temps, la question du manque d'enseignants se posera. Il faut savoir que nous utilisons déjà la télétransmission de cours- je pense notamment aux étudiants en licence professionnelle à Rodilhan, près de Nîmes, qui suivent en direct des cours dispensés depuis l'université Clermont Auvergne. Monsieur le ministre, il serait inconscient de penser que notre situation géographique suffit à elle seule à faire de la France une grande nation agricole. Cet héritage n'existerait pas sans ceux qui ont su apprivoiser nos terres. Nous devons être à la hauteur de cet héritage, et donner aux jeunes agriculteurs nécessaires à la compréhension des enjeux économiques, climatiques et même démographiques du XXI siècle. Enfin, je tiens à profiter de cette prise de parole pour souligner le formidable travail des maisons familiales rurales, celle d'Eyragues, qui doit beaucoup à l'aide que lui accorde le département-je sais que tel n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire national. En somme, monsieur le ministre, l'agriculture de demain se prépare aujourd'hui. Il s'agit de se montrer à la hauteur. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'enseignement agricole dans notre pays est exemplaire, et pourtant nous n'en parlons presque jamais. Celles et ceux qui le font ont du mal à être audibles, et cet enseignement est trop souvent le grand oublié des réflexions sur l'éducation. Je me réjouis donc que nous ayons ce débat- j'en remercie le groupe CRCE-, et j'espère que nos échanges auront un écho important en dehors de cet hémicycle, car les enjeux sont immenses. L'enseignement agricole permet une rencontre comme il n'en existe nulle part ailleurs entre enseignements général, technologique et professionnel, apprentissage, formation continue et même enseignement supérieur. Ses effectifs réduits permettent un apprentissage dans les meilleures conditions. est un lieu de prédilection pour le développement de pédagogies innovantes qui font la fierté de ce modèle français. Enfin, il offre un excellent taux d'insertion professionnelle. Aujourd'hui, l'enseignement agricole est à la croisée des chemins. Il est en première ligne face aux grands défis que notre agriculture doit relever : réussir la transition agroécologique et assurer la relève de toute une génération. Je crois que nous en sommes désormais toutes et tous convaincus : la transition agroécologique doit avoir lieu. Nous devons réussir à réinventer notre modèle agricole pour répondre aux besoins de la nécessaire transition écologique et envisager un modèle économique et alimentaire viable en accompagnant et en soutenant pleinement nos agricultrices et nos agriculteurs. Dire cela, c'est bien mais dire cela sans se pencher en profondeur sur l'enseignement agricole dans notre pays, sur la formation et sur les innovations qui naissent dans ces filières n'aurait aucun sens. Nous savons que les actrices et les acteurs qui le font vivre sont préparés à relever ce défi.

Il faut mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la relève, susciter l'envie, former les paysannes et paysans de demain, et garantir à celles et ceux qui s'en vont la possibilité de transmettre sereinement leurs exploitations. Nous ne pourrons pas relever ces défis sans un enseignement agricole de qualité.

pour les élèves. Mais, surtout, l'enseignement agricole, parce qu'il est pluriel, est frappé de plein fouet par toutes les dernières réformes de l'éducation : celles du baccalauréat, du lycée professionnel, de l'apprentissage, de la formation continue. Ces réformes, prises individuellement, ont suscité de vives inquiétudes. ne proviennent pas du ministère de l'agriculture, mais elles ne prennent pas en compte la spécificité de l'enseignement agricole. De plus, appliquées simultanément, elles sont en train de le déstabiliser en profondeur.

des formations, qui repose désormais avant tout sur le nombre de contrats signés, et plus sur le financement des « heures groupes » ni sur les subventions d'équilibre accordées par les régions.

plus importants, sont fragilisées, voire déséquilibrées. L'enseignement agricole est à un moment clé de son histoire. Sur le terrain, il est défendu avec passion par des personnes qui y croient et qui veulent voir ce modèle perdurer, mais elles n'y parviendront pas sans nous ! Reconnaissons la spécificité de l'enseignement agricole, rendons-le plus visible, donnons-nous les moyens de le préserver et de l'aider à relever les défis qui se profilent à l'horizon. l'horizon. En tant que parlementaires, nous devons porter la réflexion sur cette question cruciale. Ce soir, nous ne pourrons qu'effleurer le sujet, mais nous devons aller plus loin. C'est pourquoi je propose la mise en place d'un groupe de travail qui aura pour mission de produire un rapport parlementaire sur l'enseignement agricole dans notre pays. Très bien ! Prenons le temps de mener un travail collectif de qualité, qui ira au fond des choses, en nous appuyant sur les actrices et les acteurs de terrain qui ont beaucoup à nous apprendre. C'est ainsi que nous pourrons proposer une vision politique forte pour l'avenir de l'enseignement agricole en France ! La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, créé à l'origine pour former les agriculteurs, l'enseignement agricole a su évoluer et s'adapter aux besoins de la société. Les missions qui lui sont confiées en font un enseignement actif, réactif, innovant et ouvert. Il s'agit d'un précieux partenaire des acteurs des territoires. Pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain, il conviendra de porter un regard particulier sur l'innovation tant pédagogique que technologique et sur l'expérimentation. Les outils pédagogiques grandeur nature que sont les fermes et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles devront bénéficier des dernières technologies dans leur domaine d'activité et ainsi constituer une référence pour les apprenants et les professionnels. Des moyens humains supplémentaires doivent permettre aux exploitations et aux ateliers de mener leur mission d'expérimentation sans risquer de compromettre leurs résultats et, donc, l'équilibre financier auquel ils sont soumis. L'enseignement agricole constitue un réseau cohérent d'établissements, qui est structurant pour les territoires. Le département du Jura est un bon reflet de ce maillage territorial, avec notamment le réseau des maisons familiales rurales

pour tous les niveaux de formation, de recherche, de production, et la vente directe de produits transformés. Il n'y a que cinq Enilbio en France, dont deux se situent en Franche-Comté. Beaucoup de ces formations, qui vont du CAP au bac pro, au BTSA et aux diplômes d'ingénieur, se font en apprentissage. C'est pour l'avenir une voie en plein essor. Celle-ci permet aux jeunes d'avoir une connaissance de l'univers professionnel qui débouche sur un diplôme reconnu. Les jeunes issus de ces formations trouvent ensuite facilement un emploi, car ils sont immédiatement opérationnels. Plusieurs défis sont devant nous : l'évolution des activités traditionnelles, l'apparition de nouveaux usages dans la gestion de l'espace et des ressources, ou l'adaptation au changement climatique. Une évidence saute ici yeux, l'enseignement agricole devra prendre en compte le développement des métiers verts et intégrer le thème de l'environnement dans ses formations initiales. Nos agriculteurs sont et devront plus que jamais être compétitifs, efficaces, savoir anticiper et gérer les risques, inventer de nouveaux services, répondre aux défis environnementaux, tout en alliant performance économique, environnementale et sociale, garder les territoires ruraux attractifs. Autant d'enjeux qui devront être pris en compte dans l'enseignement agricole de demain. Cet enseignement agricole mène à de nombreux autres métiers très diversifiés qui sont à la croisée de l'agriculture, du numérique et de l'industrie, et qui répondent à la révolution du monde agricole qui est en train de s'accomplir. Monsieur le ministre, compte tenu de ces éléments, quels mécanismes de soutien et de diffusion de l'information pourriez-vous mettre en oeuvre, afin de favoriser une meilleure communication autour de la modernité et de la technicité des métiers auxquels l'enseignement agricole prépare ces étudiants ? Le public intéressé par ces formations- nous l'avons vu avec les MFR -est en train de changer. De plus en plus de jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole intègrent cet enseignement. Il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle.

Comment parviendrez-vous à concilier cet objectif avec la politique gouvernementale de suppression d'un certain nombre d'emplois dans l'enseignement public ? Pour que l'enseignement agricole se projette sereinement, il lui faut des moyens humains et financiers. J'en suis

MM. Guillaume Arnell et Antoine Karam -, est le second dispositif d'enseignement du pays avec plus de 800 établissements

L'enseignement agricole, c'est plus de 120 formations dans l'agriculture, bien sûr, mais aussi dans l'agroalimentaire, la filière forêt-bois, l'environnement, les services à la personne, sans oublier les formations générales. Je vous le

privé et une MFR de Magnanville, car je n'oublie pas combien ces MFR jouent un rôle essentiel dans la formation. L'enseignement agricole, c'est 60 % des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, 40 % de son budget, et ces deux chiffres sont en hausse depuis plusieurs années.

Deuxième constat, et non des moindres, l'enseignement agricole, ça marche ! Il permet aux jeunes de s'épanouir, d'obtenir un diplôme et, surtout, de s'insérer dans la société. Le taux de réussite aux examens est très élevé, vous le savez.

Plus de 6 % des élèves bénéficient d'un aménagement d'épreuves ; le nombre de jeunes bénéficiant d'un projet personnalisé de scolarisation a triplé entre les rentrées 2010 et 2018. Dans le même temps, le nombre d'auxiliaires de vie scolaire a été multiplié par six, et les crédits dédiés au handicap multipliés par sept : oui, l'enseignement agricole a les moyens de son ambition ! Les crédits augmenteront encore de 26

Je veux les saluer toutes et tous : les enseignants, les formateurs, les personnels administratifs et techniques, et les directeurs sont pleinement investis dans leur mission. Ils méritent d'être reconnus, encouragés et soutenus.

l'enseignement agricole ne serait rien, tout comme l'enseignement en général, ou encore la fonction publique, parfois tant décriée. La fonction publique, sans les fonctionnaires, marcherait beaucoup moins bien ! L'avenir, c'est de valoriser nos agents des chantiers statutaires et de revalorisation pour rendre leurs métiers plus attractifs.

reprenne des points forts de l'enseignement agricole : les contrôles en cours de formation, le rôle des oraux, par exemple. Concernant la question des spécialités,

Nos atouts, Mme Vérien l'a évoqué tout à l'heure, ce sont le cadre de vie, les internats, l'ouverture internationale, la capacité à concilier la pratique d'un sport et des études de haut niveau. Nous avons des champions de France, des champions d'Europe, des champions du monde dans nos lycées agricoles.

être fier. Je fais confiance aux établissements et à leur gouvernance inclusive pour optimiser l'offre de formation et leurs moyens. Ils le font sous l'autorité des directions

parce que, qu'on le veuille ou non, les jeunes sont sensibles à l'écologie. Le deuxième engagement consiste à rénover toutes les formations pour bien intégrer l'agroécologie et le bien-être animal. Le troisième engagement est d'atteindre des objectifs ambitieux pour les exploitations agricoles de nos lycées 100 % des 19 000 hectares d'exploitation de nos lycées devront être cultivés en agriculture biologique

plus d'agroécologie et de bien-être animal, mais aussi du numérique, de la communication, du management, des nouvelles technologies et- je vous le dis tranquillement -de la gestion. En effet, un jeune qui sort d'un lycée agricole doit savoir gérer son exploitation agricole : il sera certes paysan, mais aussi chef d'exploitation et chef d'entreprise.

de résolution pour le renforcement des sanctions adoptées par le Conseil européen contre des responsables des violations des droits humains au Venezuela

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de résolution que je vous présente aujourd'hui est destiné à renforcer les sanctions à l'encontre des responsables des violations des droits humains au Venezuela. Elle vise aussi à soutenir le dossier à la Cour pénale internationale, déjà cosigné par six pays, pour que les responsables de ces crimes soient effectivement condamnés. Je souhaite exprimer toute ma gratitude au président Hervé Marseille pour le groupe Union Centriste, au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants, ainsi qu'à tous ceux qui ont soutenu ce projet

Défenseur des droits humains, prix Sakharov 2017, M. Saleh nous a décrit les traitements inhumains auxquels il a été soumis lors de son emprisonnement dans une cellule de torture appelée « la tombe ».

Au Venezuela, être un opposant politique implique un prix très lourd à payer : en 2019, plus de 50 manifestants ont été abattus par les forces de l'ordre ou par les, des ou par les, des groupes paramilitaires terrorisant et contrôlant la population et qui, bien sûr, sont aux ordres du régime Maduro. Dans ce pays, la violence est une politique d'État. 18 000 personnes ont été tuées depuis 2016 selon l'ONU, pour qui il s'agit d'un « modèle de conduite systématique Vous avez tous reçu hier, mes chers collègues, une lettre du représentant de Nicolás Maduro en France, lequel assure que son pays est accusé d'assassinats sans preuve. C'est le propre des régimes criminels de ne pas se confronter à leurs actes et de nourrir le négationnisme ! Le rapport très documenté de la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, publié le 4 juillet dernier, dénonce un « nombre extrêmement élevé » d'exécutions extrajudiciaires. Entre le moment où nous commençons ce débat et celui où nous le conclurons, il y aura 2 morts assassinés pour « résistance à l'autorité ». Il s'agit de femmes et d'hommes comme ce conseiller municipal, Fernando Albán, jeté d'un dixième étage par le service d'intelligence militaire du régime.

torturé, assassiné, son corps calciné abandonné. Quelle horreur ! Et cela au moment même où le Venezuela obtenait un siège au Conseil des droits de l'homme des Le crime de M. Rada ? Être un leader politique apprécié à Petare, le- bidonville -le plus important du pays. Personne ne doit ignorer que Nicolás Maduro et ses appuis militaires persécutent, font disparaître et massacrent la population vénézuélienne. Le Venezuela est le premier pays d'Amérique latine où je me suis rendu, voilà quatre ans. Il est connu comme le pays disposant des réserves pétrolières les plus importantes au monde. pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, les réserves prouvées de ce pays atteindraient les 297 milliards de barils, le plaçant à la première place mondiale devant l'Arabie saoudite. Mais ce pays est aussi celui des records pour l'inflation,

Cette crise a déclenché une situation d'urgence humanitaire complexe, à laquelle personne n'échappe. Les Vénézuéliens subissent de graves pénuries d'eau et de médicaments. Au moins 80 % de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Pourquoi le Venezuela, ce pays si riche, est-il devenu aussi pauvre ? La raison principale est que le système du chavisme est fondé sur une corruption endémique ayant rongé tous les corps de l'État. Le régime de Nicolás Maduro pourrait nous paraître à bout de souffle. Mais ne nous trompons pas ! Si le chavisme tient encore, c'est notamment grâce à l'exploitation illégale des ressources présentes dans l'Amazonie, dans une zone connue comme l'. Cette zone est un atout sans égal pour le régime. Elle comporte des réserves exceptionnelles en or, diamant, cuivre, fer et coltan. Elle couvre une superficie de 112 000 kilomètres carrés et représente l'oxygène nécessaire pour le régime. L'exploitation des minéraux dans l'n'est pas sans conséquence pour l'environnement, avec le déversement colossal de produits toxiques comme le cyanure et le mercure, les populations indigènes, qui sont spoliées de leurs terres, exploitées et font l'objet de toutes formes de violences. Vous l'avez bien compris, mes chers collègues, le Venezuela est un État failli. est un État failli. C'est un État où des groupes criminels font partie des forces de l'ordre. C'est un territoire où les groupes terroristes opèrent librement. C'est un État qui entretient des liens étroits avec la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba ... autant d'États dont le soutien est animé par des raisons géopolitiques et, disons-le franchement, peu regardants en matière de droits humains. Le pouvoir chaviste a détruit le cadre institutionnel, mis à bas le secteur privé et soumis la population pour piller librement les ressources du pays. En vingt ans de chavisme, 393 milliards d'euros d'actifs issus de faits de corruption sont sortis du Venezuela selon la commission des finances du parlement vénézuélien. Dans le même temps, le pays vit la pire crise humanitaire de son histoire et les Vénézuéliens partent massivement à cause de cette situation. Chaque jour, 5 000 personnes traversent la frontière à la recherche d'une vie digne. Plus de 4,5 millions de personnes sont déjà réfugiées dans les pays environnants. D'ici à 2020, environ 8 millions de Vénézuéliens auront quitté leur pays. Ce chiffre est supérieur au nombre de personnes ayant quitté la Syrie en guerre ! C'est une crise de portée régionale qui affecte désormais tous les pays du continent. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. La France, aussi, doit montrer aux Vénézuéliens qu'ils ne sont pas seuls. Nous avons un devoir à l'égard de ces populations. Nous souhaitons entretenir l'espoir de jours meilleurs. La France est une puissance de paix. Elle soutient toutes les médiations pour sortir de ce drame par une voie politique. Je veux remercier le Gouvernement, madame la secrétaire d'État, d'avoir fait ce choix. Je souhaite aussi saluer l'action exemplaire de Romain Nadal, notre ambassadeur au Venezuela, et de toute l'équipe du poste diplomatique à Caracas, qui oeuvre au quotidien aux côtés des artisans d'une solution politique pour le Venezuela. Mais la France, c'est aussi le berceau des droits de l'homme. Ceux qui tirent avantage du régime dictatorial de Maduro ne doivent pas pouvoir en vivre impunément sur notre sol. La France ne saurait être un sanctuaire pour eux C'est pourquoi nous proposons cette résolution pour le renforcement des sanctions contre les responsables des violations des droits humains au Venezuela et pour soutenir les pays signataires de l'enquête auprès de la Cour pénale internationale. À travers ce document, nous appelons les autorités françaises à être vigilantes quant aux fonds provenant du Venezuela et, plus particulièrement, ceux des responsables sanctionnés par l'Union européenne, rappelant que les sanctions prises par cette dernière devront être appliquées dans tout l'espace Schengen, et donc en France. De même, nous appelons les autorités à être vigilantes quant aux possibles liens avec le trafic de drogue ou le terrorisme. En dernier lieu, nous appelons la France à rejoindre les pays signataires du dossier en cours devant la Cour pénale internationale et à soutenir son procureur, Mme Fatou Bensouda, afin que les responsables des violations des droits de l'homme afin que les responsables des violations des droits de l'homme soient condamnés. Pour finir, en saluant la présence dans la tribune de Mme Isadora Zubillaga, représentante en France du président par intérim Juan Guaidó, je tiens répéter combien il est important de soutenir le peuple vénézuélien par cette démarche.

la secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sociale, économique et politique au Venezuela est grave. Elle laissera des traces dans le pays pendant de longues années. Personne n'est insensible à cette situation, surtout pas nous. Mais la proposition de résolution qui nous est soumise est-elle la contribution attendue de la France face à une telle situation ? Nous ne le pensons pas

de résolution invitent en effet le Sénat à emboîter le pas, sans nuance, à ceux qui reconnaissent Juan Guaidó comme président autoproclamé, alors même que son soutien à l'intérieur du pays recule fortement au rythme des révélations des révélations sur ses liens directs avec les entreprises de déstabilisation engagées sur l'initiative des États-Unis. Ces mêmes attendus mettent en cause la Russie, avec une rhétorique de guerre froide qui conduira, une fois de plus, la France à se marginaliser dans la région si nous en suivions le fil. Je crois qu'il y a bien mieux à faire ! La situation de crise est grave, je l'ai dit. La crise politique est devenue une crise violente. Les Vénézuéliens en paient un prix élevé. aujourd'hui de 3,7 millions de Vénézuéliens ayant quitté le pays et 80 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les causes de la crise sont multiples. Après des années de lutte contre les inégalités et la pauvreté financées par la manne pétrolière, l'affaissement des cours du pétrole a replongé le pays dans d'importantes difficultés, faisant reculer le PIB de 50 % depuis 2015. Ce recul brutal a d'autant plus déstabilisé l'économie nationale en termes de stratégie économique n'ont pas toujours été appropriées. Ces erreurs sont d'ailleurs débattues au sein même des forces qui soutiennent Nicolás Maduro et refusent la prise de pouvoir de Juan Mais il est clair, et les attendus de la proposition de résolution n'en disent rien, bien au contraire, que cette déstabilisation a été souhaitée et clairement alimentée par les États-Unis, qui ont saisi là l'occasion, après la mort d'Hugo Chávez, d'en finir avec une expérience politique dont ils n'ont jamais voulu.

Pourquoi le nier quand Donald Trump, lui-même, s'en vante ? Et pourquoi s'en tenir à emboîter le pas à la rhétorique américaine sans prendre aucun recul ? Pour les États-Unis, le Venezuela est une clé de voûte en Amérique latine, où, en même temps, ils renforcent les sanctions illégales contre Cuba, soutiennent de toutes leurs forces le régime de Jair Bolsonaro, appuient les gouvernements du Chili et de l'Équateur réprimant les révoltes populaires. Est-ce l'intérêt de la France de suivre cette doctrine qui fleure bon le retour de la « doctrine Monroe » en Amérique latine ? Le Venezuela a surtout besoin d'un retour à la stabilité politique, à la paix, à la réconciliation pour retrouver le chemin du développement. Et il a besoin pour cela d'un plein respect de sa souveraineté et d'un processus politique négocié de sortie de crise.

les autres par l'opposition. Sortir de cette situation par la violence, voire, pire, par la guerre civile dont le spectre plane, serait un calcul effroyable. La droite vénézuélienne a sa responsabilité dans l'engrenage des violences. Les trois gouverneurs qu'elle a fait élire dans le bassin du lac de Maracaibo, le long de la frontière colombienne, l'ont été dans une région où le pouvoir du crime organisé est évident, tout comme l'implantation de longue date des narcotrafiquants et des paramilitaires.

le retour des députés de la majorité présidentielle au sein de l'Assemblée nationale vénézuélienne, à la suite d'un accord avec une partie importante de l'opposition, est un premier pas à saluer. La France devrait appuyer le Mexique et l'Uruguay, qui ont proposé leur médiation, et les efforts de la Norvège pour ouvrir à Oslo un dialogue entre le président Maduro et les forces d'opposition de l'assemblée vénézuélienne. La France devrait entendre l'appel de l'ONU mettant en garde contre les conséquences des mesures coercitives unilatérales en ces termes : « Ce n'est pas la réponse à la situation politique du Venezuela. » Cet appel souligne « l'urgente nécessité pour tous les acteurs concernés de participer à un dialogue politique inclusif et crédible pour aborder la longue crise que traverse le pays, dans le plein respect de l'État de droit et des droits humains ». Évidemment, la situation des droits humains est au coeur des enjeux de la sortie de crise. Le rapport de Michelle Bachelet pour l'ONU chiffre à 5 000 le nombre de personnes tuées par les forces de sécurité en 2018, dans la spirale de violences alors provoquée. Près de 400 fonctionnaires des Forces d'action spéciales sont actuellement jugés pour ces délits. Il faut se féliciter que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ait signé un accord avec le Venezuela pour renforcer leur coopération, avec l'objectif d'ouvrir un bureau permanent sur place. Deux représentants de l'ONU sont autorisés à rester et à accéder à tous les centres de détention. À l'opposé des sanctions décidées par Washington et soutenues par la présente proposition de résolution, nous devrions donc soutenir les efforts de dialogue, d'où qu'ils viennent, et associer la France à ces efforts. Cette proposition est à contre-courant de cette ambition. Elle se contente d'alimenter un portrait caricatural d'une situation particulièrement complexe. C'est pourquoi nous voterons contre ce texte. C'est dommage ! La parole est à M. Alain Fouché.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nombreux sont les rêves d'inspiration marxiste ou communiste qui ont tourné et tournent encore au cauchemar. L'un d'entre eux s'annonce particulièrement long et douloureux. Près de 15 % de la population a fui le pays ... Au sein de ceux qui restent, cela a été dit, 94 % vivent sous le seuil de pauvreté ... Bienvenue à Caracas ! Le pays ne parvient pas à sortir de la crise qui a dégénéré lorsque Nicolás Maduro a proclamé sa réélection, à l'issue d'un scrutin truqué. suite de cette fraude électorale, dénoncée dans le monde entier, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, a été reconnu président par intérim par 55 pays,

Il a néanmoins surpris par le degré de violence employé pour se maintenir en place. L'ONU dénonce l'usage systématique d'une « force excessive » à l'encontre des manifestants. Cet euphémisme est bien pudique quand, depuis 2018, plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées, torturées, assassinées. Et cela continue

Pour tenter de sortir de la crise, la communauté internationale avait deux choix : ne rien faire ou intervenir. Plusieurs pays soutiennent le régime en place,

Dormez tranquilles, braves gens, l'équipe de choc de la démocratie est au chevet du Venezuela ! oubliant, dans un délire de révolutionnaire de salon, que, si lui-même avait été un opposant politique au Venezuela, il aurait peut-être été défenestré du dixième étage par les forces de sécurité, comme le fut Fernando Albán. En janvier, puis en août, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions au régime. Ils imaginent, comme dans le dossier iranien, que cela poussera la population ou l'armée à renverser le pouvoir en place. Mais pour l'heure : beaucoup de tweets, pas de résultat ! Le Conseil européen a lui aussi infligé des sanctions au régime. Certains dénoncent l'emploi de telles sanctions, au motif qu'elles aggravent la crise humanitaire. Mais quelle est l'alternative ? Ne rien faire et laisser ce peuple sombrer chaque jour un peu plus dans la misère et dans la torture ? Nous sommes convaincus que les Vénézuéliens doivent pouvoir choisir librement leurs dirigeants. Il nous semble que l'emploi de la force n'est pas ce dont le pays a besoin. La sortie de la crise ne pourra être que politique nous croyons que les sanctions économiques contre le régime vont l'inciter à négocier. En parallèle, il nous faut agir pour protéger la population, pour protéger le règne de la loi. Les atteintes aux droits de l'homme doivent cesser. Le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête préliminaire en 2018 pour violations des droits humains et crimes contre l'humanité. Sans justice, la paix ne pourra pas revenir au Venezuela. L'action de la Cour pénale internationale prendra, hélas, du temps- c'est toujours long -, mais on ne peut que la soutenir. Nous avons été nombreux à signer cette proposition de résolution, qui se justifie pleinement tant ce peuple est maltraité et vit dans des conditions scandaleuses. Je ne comprends pas que l'on puisse y être opposé. Nous ne pouvons rien faire de mieux que d'imposer des sanctions économiques. Les Européens doivent s'interroger sur la stratégie à mettre en oeuvre, d'une manière générale et quelles que soient leurs tendances, face aux régimes autoritaires. Le groupe auquel j'appartiens,

Syrie, Sahel, détroit d'Ormuz, Corée du Nord, Algérie, Liban, Chili : les foyers de crise et d'inquiétude sont, ces derniers temps, si nombreux et si complexes sur la scène internationale qu'on en aurait presque tendance à oublier un peu rapidement ceux qui ne font pas quotidiennement les gros titres des journaux. Cette proposition de résolution, présentée par notre excellent collègue Olivier Cadic, a donc pour mérite de remettre sur le devant de la scène le Venezuela, et l'état catastrophique dans lequel ce pays se trouve depuis maintenant plusieurs mois. Si le monde s'en était légitimement ému et alerté au plus fort des tensions politiques, l'enlisement de la situation nous a malheureusement presque fait « passer à autre chose ». Or c'est pour cette raison même qu'il n'a jamais été aussi urgent de venir en aide à ce pays et à sa population. Alors que le Venezuela fut longtemps la nation la plus prospère et la plus développée d'Amérique latine, et Caracas la perle du continent, il est aujourd'hui le théâtre d'une crise humanitaire sans précédent dans un pays ayant atteint un tel niveau de développement. triste démonstration de la « malédiction des ressources naturelles » que nous offre ce pays, qui a détruit son économie en la soumettant entièrement aux lois du cours du baril de pétrole. Alors que crise politique et crise économique se nourrissent l'une l'autre depuis maintenant des années, des vents contradictoires soufflés par la communauté internationale viennent attiser les braises. Quelle ironie de voir que la crise traversée par le Venezuela a réactivé de vieux clivages stratégiques que l'on croyait disparus depuis les années 1990 En effet, alors que Juan Guaidó est reconnu par le Groupe de Lima, les États-Unis et la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, les principaux piliers extérieurs du régime de Maduro ne sont autres que la Chine, la Russie, la Turquie, l'Iran, le Nicaragua et Cuba.

Près de 10 % de la population vénézuélienne a en effet émigré vers les pays voisins, ne supportant plus le manque de médicaments, les coupures d'eau et d'électricité, l'inflation à 1 000 000 % et l'insécurité croissante. Ces migrants Ces migrants se sont majoritairement déplacés vers les pays voisins, au premier rang desquels la Colombie, ce qui fait peser un poids dramatique sur leurs épaules. La France n'est pas restée inactive, encore moins indifférente, depuis le début des difficultés du régime de Maduro. En effet, alors que la relation franco-vénézuélienne s'était dégradée depuis 2017, dans le contexte d'attaques verbales de Nicolás Maduro, nous avons durci notre position à son égard. En 2018, la France a apporté son soutien à la demande adressée à la Cour pénale internationale par cinq États latino-américains et le Canada, afin d'ouvrir une enquête sur les accusations de crimes contre l'humanité visant le régime de Nicolás Maduro, demande à laquelle la Cour pénale a répondu favorablement le 8 février 2018. Un examen préliminaire de la situation est en cours, et nous serons bien entendu très attentifs aux conclusions Enfin, notre pays a reconnu Juan Guaidó comme « président en charge » pour mettre en oeuvre un processus électoral dès le 4 février 2019. Par ailleurs, la France a apporté une aide humanitaire importante au Venezuela et aux pays voisins touchés par la crise migratoire. L'Europe n'a pas non plus gardé les bras croisés, et ce malgré l'absence d'un consensus absolu de ses membres pour la reconnaissance de la légitimité présidentielle de Juan Guaidó. J'en veux pour preuve la conférence internationale qui s'est achevée hier à Bruxelles, sous l'égide du Service européen pour l'action extérieure, le SEAE, et qui a tenté d'apporter des réponses à la crise des réfugiés qui qui fait rage. Cette proposition de résolution va résolument dans le bon sens : il apparaît effectivement important d'être vigilant quant aux fonds provenant du Venezuela et de veiller à appliquer les sanctions et les limitations décidées. Je m'attarderai plus particulièrement sur la dernière de ces recommandations : faire en sorte que l'État français rejoigne les pays signataires du dossier en cours auprès de la Cour pénale internationale et soutienne le procureur, Mme Fatou Bensouda, pour que les responsables des violations des droits humains soient condamnés. Signe, s'il en fallait un, de la gravité de la situation, ce sont pour la première fois des États, et non des individus, qui formulent contre un autre État une plainte auprès de la Cour pénale internationale de La Haye. Si la France a déclaré soutenir cette initiative, elle n'a pas pour autant rejoint les six pays signataires de la plainte. Pourquoi donc, madame la secrétaire

La crise humanitaire est aiguë. La quasi-totalité de la population de ce pays, autrefois si riche, vit aujourd'hui dans la pauvreté, voire dans l'extrême pauvreté. Les pénuries de nourriture, les difficultés d'accès aux soins et aux médicaments, les coupures d'électricité, le délabrement des infrastructures publiques rendent la vie insupportable. Il ne s'agit d'ailleurs plus de vivre, mais de survivre. Au total, 7 millions de Vénézuéliens ont besoin d'aide humanitaire et, dans le pays, près d'un quart des enfants souffrent de malnutrition. cette situation est d'abord le résultat d'une gestion catastrophique du pays, d'un manque d'investissements et d'une corruption aggravée qui durent depuis des années. Dans ce contexte épouvantable,

pays. Cet exode sans précédent fait courir de nombreux dangers aux personnes qui prennent la route- parfois des mineurs isolés -, livrées aux passeurs, victimes des réseaux de traite, condamnées à vivre dans la rue, dans les villes où elles atterrissent.

Mais le régime fait tout pour entraver les secours. En effet, cette grave crise a évidemment un volet politique. Depuis 2018, le Parlement démocratiquement élu est privé de ses pouvoirs, les médias sont entravés les contre-pouvoirs démantelés. En plus des privations qu'ils supportent au quotidien, les Vénézuéliens subissent une féroce répression de la part du régime, qui veut étouffer tout mouvement de protestation arrestations arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, la torture sont couramment pratiquées, y compris sur des représentants du peuple démocratiquement élus. Selon le gouvernement chaviste lui-même, plus de 1 500 personnes auraient été tuées lors d'opérations de sécurité durant les six premiers mois de l'année 2019. Près de 800 personnes seraient détenues arbitrairement ; on ne compte plus les rapports qui témoignent des graves violations des droits de l'homme et des atteintes à l'État de droit commises dans ce pays.

La solution à la crise ne peut qu'être politique. Malheureusement, nous ne voyons aucun signe d'espoir. Les tentatives de médiation entre le régime et l'opposition, que ce soit celle d'Oslo ou celle menée dans le cadre du groupe international de contact, le GIC, sont au point mort. Le régime Maduro se borne à un simulacre de dialogue avec l'opposition minoritaire. La « feuille de route » prévoit la tenue d'élections législatives, mais le calendrier reste plus qu'incertain. Pour sortir de l'impasse politique actuelle, c'est une élection présidentielle libre et transparente, dans le cadre d'une transition négociée, qui serait nécessaire. Il s'agit là d'une condition au rétablissement de la démocratie et de l'État de droit au Venezuela. la France et par l'Union européenne, dont vingt-quatre États membres reconnaissent le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, président par intérim, mais il est refusé par le régime chaviste. L'impasse politique ne peut que pousser la population désespérée à reprendre le chemin de la rue. Dans ce contexte, il faut soutenir les initiatives récentes prises à l'échelle européenne pour renforcer les mesures restrictives à l'encontre du régime chaviste. chaviste. Ainsi, le 25 septembre dernier, des sanctions individuelles ont été imposées contre 7 membres des forces de sécurité accusés de torture. Cette décision porte à 25 le nombre de responsables vénézuéliens visés par des interdictions de visas et des gels d'avoirs dans l'Union européenne. proposition de résolution appellent nos autorités à une application stricte de ces sanctions ainsi qu'à une vigilance particulière à l'égard des fonds provenant du Venezuela : leur origine peut être douteuse compte tenu des organisations criminelles qui prospèrent dans le pays. En outre, ils invitent la France à rejoindre les pays ayant engagé une procédure auprès de la Cour pénale internationale sur les accusations de crime contre l'humanité prononcées contre le régime de Nicolás Maduro Moros. Pour l'heure, notre pays ne fait que soutenir la demande formulée par d'autres États, à savoir cinq pays latino-américains et le Canada. Certes, une procédure devant la CPI est nécessairement longue. Mais, plus que le résultat, c'est ici le message qui compte : cette procédure signifie d'abord la reconnaissance, par la communauté internationale, du drame vécu par des millions de Vénézuéliens,

fort. Le président vénézuélien continue d'opprimer son peuple. Il ne manifeste aucun signe de faiblesse : au contraire, il se mêle d'apporter son soutien aux mouvements de contestation qui secouent actuellement l'Équateur et le Chili.

La crise que connaît le Venezuela a éclaté il y a maintenant six ans, avec la mort d'Hugo Chávez et la désignation de son successeur Nicolás Maduro. La contestation de la légitimité de cet héritier a pris une dimension supplémentaire en 2015, lorsque l'opposition a remporté les élections législatives. Elle a conduit à un démantèlement des contre-pouvoirs et à une remise en cause de l'État de droit. Le 23 janvier 2019, Juan Guaidó, président d'une Assemblée nationale vidée de ses pouvoirs et prérogatives, s'est autoproclamé président par intérim. Il a été reconnu par de nombreux États-

entre novembre 2018 et février 2019, on a compté 1 557 personnes décédées en raison de l'approvisionnement défectueux des hôpitaux.

Des députés de l'opposition sont poursuivis malgré leur immunité parlementaire, contraints de fuir ou de se réfugier dans des ambassades étrangères. Les manifestations sont réprimées brutalement : chacun a pu le constater. Selon le rapport du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme du 4 juillet 2019, 793 personnes sont arbitrairement privées de leur liberté, et 66 autres seraient décédées lors des manifestations qui se tiennent depuis janvier 2019. Le gouvernement vénézuélien lui-même-

miser sur le renversement du président Maduro par une population le considérant comme responsable de sa situation économique et sociale. Mais le pari semble perdu le régime Maduro reste en place. Il dispose encore du soutien de l'armée et- d'autres l'ont dit avant moi -de certaines puissances internationales. Il y a, de l'autre côté, le choix des Européens

nous sommes face à un régime qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête internationale pour violation des droits humains et fait fi des règles élémentaires de tout État de droit, de toute démocratie : il doit être condamné, et nous le condamnons.

le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a décidé, le 27 septembre dernier, l'ouverture d'une enquête par une mission internationale indépendante sur les violations des droits humains au Venezuela depuis 2014. Cette demande avait été formulée, dès 2018, par cinq États d'Amérique latine et par

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la situation politique au Venezuela suscite de vives inquiétudes, tant elle réveille le souvenir d'une époque tragique, celle des « années de plomb » qu'avaient subies de nombreux pays d'Amérique latine au cours des décennies 1960 et 1970. Alors que Caracas s'était démarquée en entamant dès 1958 une longue tradition démocratique, le régime actuel est accusé d'abuser de pratiques totalitaires que l'on espérait révolues sur le continent sud-américain. Nous connaissons les conditions troubles dans lesquelles Nicolás Maduro a été réélu en 2018. Certains orateurs les ont rappelées. La France les a déplorées et c'est une bonne chose : le dirigeant vénézuélien a choisi non seulement de tourner le dos à la démocratie, mais aussi d'entrer en conflit ouvert avec une partie significative de sa population. Amnesty International et le Conseil des droits de l'homme des Nations unies ont respectivement dressé un bilan sans appel des violences commises depuis 2014 au Venezuela : plus de 14 000 personnes auraient été arrêtées de façon arbitraire sous le motif officiel de « résistance à l'autorité » ; des centaines d'exécutions extrajudiciaires auraient été perpétrées en pleine rue les manifestations seraient réprimées et les opposants torturés par les forces armées spéciales, les FAES, créées en 2017. Le climat intérieur est d'une telle violence que de nombreux Vénézuéliens choisissent l'exil. En cinq ans, plus de 4 millions de personnes ont officiellement quitté le pays. En accueillant 1,5 million de réfugiés, la Colombie a largement ouvert ses frontières, mais la coopération entre pays voisins commence à se dégrader. Depuis l'été dernier, de peur d'être déstabilisés dans un contexte économique régional difficile, le Pérou, le Chili et l'Équateur ont entrepris de durcir leurs conditions d'entrées.

nos territoires d'outre-mer présents dans cette aire géographique pourraient être affectés. C'est d'ailleurs déjà le cas de mon territoire, Saint-Martin, par ailleurs fragilisé par l'ouragan Irma. soyons attentifs à ce qui se passe en Bolivie, avec la victoire contestée d'Evo Morales dimanche dernier. Madame la secrétaire d'État, je sais que le Gouvernement est parfaitement mobilisé sur ce dossier sensible, à l'instar de l'Union européenne. Bien entendu, les élus du RDSE soutiennent toutes vos initiatives destinées à encourager la reprise du dialogue entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition, ainsi que celles visant au rétablissement des libertés fondamentales. nous nous inquiétons des moyens de pression limités dont dispose la communauté internationale, surtout quand la Chine et la Russie, une fois de plus, Tout d'abord- vous le savez, mes chers collègues -, la souveraineté des États étant protégée en droit international, toute ingérence directe doit être évitée.

En effet, le Venezuela est entré au Conseil des droits de l'homme de l'organisation, pour la période 2020-2022, alors que ce même conseil a diligenté, en septembre 2019, une mission d'enquête sur la violation des droits de l'homme doit nous amener à nous interroger sur le fonctionnement des institutions multilatérales. Ces dernières ont besoin d'un minimum de crédibilité pour être efficaces, de surcroît dans un contexte où elles sont de plus en plus contestées. Pour autant, il est utile de rappeler que le Venezuela a des engagements internationaux à honorer, en particulier la convention contre la torture, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'intervention militaire est inenvisageable

Le RDSE soutient cette demande, tout en gardant à l'esprit que les sanctions internationales n'ont pas toujours non plus la portée que l'on souhaiterait, n'en déplaise au président Wilson, qui déclarait en son temps qu'« une nation boycottée est une nation en voie de capitulation » et que ce remède « pacifique et silencieux » évitait le « recours à la force ». Le cas de l'Irak démontre qu'un pays peut être atteint par le plus dur régime de sanctions sans être pour autant épargné par une intervention militaire. Plus généralement, les sanctions font rarement plier un régime. L'Iran, la Corée du Nord et la Russie, laquelle a été visée après l'annexion de la Crimée, se sont à peine émus de leur situation ! Madame la secrétaire d'État, sans relâcher les efforts diplomatiques pour tenter d'isoler le régime de Nicolás Maduro, nous avons donc la responsabilité d'apporter une aide humanitaire à tous les Vénézuéliens qui sont en danger. Nos collègues appellent à une action vigoureuse de la part de la Cour pénale internationale. Les Vénézuéliens ne trouveront pas justice dans leur pays, c'est certain au sommet de l'État figure le Tribunal suprême de justice, une institution dominée par des proches de l'exécutif. Justice doit donc leur être apportée à l'extérieur. du RDSE voteront cette proposition de résolution, car le respect des droits de l'homme a toujours été au coeur des actions de la France sur la scène internationale. Nos amis vénézuéliens appellent au secours. Malgré les difficultés que j'ai évoquées, le renoncement n'est pas dans les gènes de notre République. Vous pouvez donc être assurés du soutien de mes collègues du RDSE et de moi-même, pour les nouvelles initiatives que la France engagerait et qui donneraient un peu d'espoir au peuple vénézuélien,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Venezuela est, depuis six ans, le théâtre d'une crise économique effroyable, d'un désastre humanitaire et de troubles politiques assortis de violations massives des droits humains, responsables d'une migration sans précédent.

avec la force publique. Plus de 4 millions de Vénézuéliens ont fui leur pays et, à l'intérieur, l'exode provoqué par l'insécurité et les déplacements forcés de population est encore plus massif. De nombreux témoignages ont permis d'établir qu'une grande majorité de ces violences est le fait des forces de sécurité fidèles au président déchu. Les opposants politiques sont, eux aussi, la cible d'attaques en règle, menées au mépris des immunités parlementaires. Les auteurs de ces violences et attaques jouissent d'une impunité totale aucune enquête judiciaire sérieuse n'a été diligentée. Aussi, la démocratie et l'État de droit ne seront possibles au Venezuela que si l'on arrive à une solution politique du conflit. Celle-ci passe par un dialogue, selon des règles clairement établies, intégrant tous les courants politiques, notamment ceux qui rejettent la violence. Or Nicolás Maduro est décidé à gouverner seul. Différents subterfuges ont été employés, dont le plus significatif est la mise en oeuvre inconstitutionnelle d'une assemblée constituante de citoyens. Cette dernière tactique avait pour seul but de déposséder de son pouvoir législatif le Parlement, alors dominé par l'opposition. C'est dans ce contexte, en dehors du cadre constitutionnel, que s'est déroulée l'élection présidentielle de 2018, boycottée par l'opposition et dont Nicolás Maduro se prévaut. Dès lors, en l'absence de président légalement élu et conformément à la Constitution vénézuélienne, il est revenu au président de l'Assemblée nationale, Juan Guaidó, d'assurer les fonctions de président par intérim à titre provisoire, le temps que des élections libres et démocratiques soient organisées dans un délai de trente jours. La France, les États-Unis et une partie de la communauté internationale n'ont fait que reconnaître une situation qui a découlé de l'application même de la Constitution du Venezuela. Nous n'avons fait que reconnaître la volonté du peuple vénézuélien telle qu'elle est exprimée dans sa loi fondamentale. Jouant, depuis lors, sur les divisions partisanes, les héritiers de Chávez ont ajouté à la confusion la terreur, créé la pénurie alimentaire et la précarité énergétique, finissant de dilapider la manne pétrolière. Ils ont même poussé le cynisme jusqu'à revendiquer un poste au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, fragilisant encore un peu plus la crédibilité de ce conseil. Sans préjuger d'autres initiatives, la France a d'ores et déjà plaidé pour la mise en oeuvre d'un processus électoral démocratique et pacifique, sous la conduite du seul dirigeant légitime du Venezuela, Juan Guaidó. soutenu la Cour pénale internationale dans l'interpellation et le jugement des partisans de Maduro, soupçonnés d'être responsables ou complices de graves violations des droits de l'homme.

Celui-ci ressemble de plus en plus à une expérience transformant les Vénézuéliens en cobayes d'une dictature populiste où les adversaires politiques sont considérés comme des ennemis du peuple. Regardons les choses en face ! Le régime de Maduro s'est changé en un pouvoir autoritaire et agressif, incompétent et corrompu.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes, comme vous, très préoccupés par la situation du Venezuela.

Depuis le premier semestre de l'année 2019, le nombre de personnes en besoin d'assistance alimentaire a quasiment doublé et représente désormais 10 millions à 14 millions de personnes, selon les chiffres du groupe de contact international auquel la France participe. Ces chiffres n'incluent pas les 4,3 millions de Vénézuéliens qui ont déjà quitté leur pays. L'exode en cours pourrait concerner 7 millions de personnes d'ici à la fin de l'année 2020, ce qui constitue la seconde crise migratoire à l'échelle mondiale, derrière la Syrie, mettant sous pression les infrastructures d'accueil de tous les États de la région. Face à ce constat, il est essentiel de permettre l'accès des acteurs humanitaires au territoire vénézuélien. Sur le plan politique, nous sommes confrontés à un blocage des discussions qui devaient aboutir à la mise en place d'un processus électoral libre et crédible. Le processus de médiation dit d'Oslo entre le régime et l'opposition a été ajourné le 15 septembre par l'opposition, après que M. Maduro a lui-même suspendu, au mois d'août, sa participation à cet espace de dialogue. Alors, face à l'impasse, la France et l'Union européenne portent le même message. L'issue à cette crise ne peut être que pacifique et négociée. Elle passe par l'organisation d'élections présidentielles crédibles qui permettront au peuple vénézuélien de choisir de nouveau son destin. Le groupe de contact international, auquel participe la France, a pour mandat de créer les conditions d'une telle solution négociée, tout en améliorant l'accès de l'aide humanitaire aux Vénézuéliens. Ce groupe de contact, qui s'est encore réuni cette semaine, a permis des progrès significatifs en matière d'acheminement de l'aide humanitaire. Sur le plan politique, ce groupe appelle à la tenue, dès que possible, d'élections présidentielles libres, transparentes et crédibles. Il incite à travailler, pour y parvenir, à l'élaboration d'une feuille de route recensant les garanties nécessaires à mettre en oeuvre pour y arriver. Le groupe de contact international constitue aujourd'hui le seul groupe capable de parler aux deux parties. Ces efforts coordonnés doivent être poursuivis et encouragés, et vous pouvez compter sur nous pour ce faire. Par ailleurs, nous rejetons fermement tout recours à la force, qu'il soit le fait des Vénézuéliens eux-mêmes ou de puissances étrangères. Pendant que les discussions sont suspendues, les droits de l'homme sont toujours bafoués par le régime de Nicolás Maduro, comme l'a tristement documenté le rapport publié le 5 juillet dernier par la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies, Mme Michelle Bachelet. La répression touche avant tout les populations les plus défavorisées et de fortes présomptions d'exécutions extrajudiciaires dans les quartiers populaires ont été mises en lumière par la haut-commissaire. Je tiens à le dire ici très solennellement, la France appuie sans réserve l'action de la haut-commissaire et condamne fermement la répression violente des manifestations, ainsi que les menaces et les violations des droits de l'homme survenues dans les derniers mois à l'encontre d'élus

Nous appelons également à la libération immédiate, complète et irréversible des prisonniers politiques. Ces violations des droits de l'homme nous conduisent à regretter que le Venezuela ait été élu, il y a deux semaines, par l'Assemblée générale des Nations unies pour siéger pendant trois ans au Conseil des droits de l'homme. La France, en lien avec ses partenaires européens, veillera avec rigueur à la manière dont le Conseil conduira sa mission l'an prochain dans ce contexte, comme l'a indiqué, dès le 22 octobre dernier, la porte-parole de Federica Mogherini, la Haute Représentante de l'Union européenne.

J'en viens aux différentes questions et remarques au coeur de cette résolution sur les initiatives actuellement prises par la France pour faire cesser les atteintes aux droits de l'homme au Venezuela. Tout d'abord, votre résolution nous interroge sur notre position à l'égard de l'enquête préliminaire de la Cour pénale internationale concernant le Venezuela. La position de la France ne varie pas : nous soutenons, sans réserve, sans préjugé, sans arrière-pensée, la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, considérant qu'elle contribue directement à la paix, à la stabilité et à la sécurité internationales tout en répondant à une demande de justice légitime de la part des victimes. En septembre 2018, le Canada et cinq États latino-américains- Argentine, Chili, Colombie, Paraguay et Pérou -ont adressé à la Cour pénale internationale un renvoi concernant la situation au Venezuela depuis février 2014 et demandant au procureur d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes contre l'humanité. Le Président de la République s'est exprimé clairement sur ce sujet : le processus en cours concernant le Venezuela est bien de nature à établir les faits qui ont conduit à la crise et à contribuer ainsi à y trouver une issue. c'est la première fois depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome en 2002 qu'un groupe d'États défère une situation concernant le territoire d'un autre État partie, également lié par ce statut devant la Cour pénale internationale. Au-delà du cas précis du Venezuela, cette appropriation nouvelle du statut de Rome montre l'importance du rôle de cette Cour pénale internationale et la promotion, par de nombreux États, de la lutte contre l'impunité. Nous suivons donc avec attention la procédure actuellement menée par le bureau du procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, qui étudie l'ouverture d'une enquête. Notre position consiste à soutenir les travaux de la CPI et à faire une confiance totale, sans réserve et sans arrière-pensée, à cet organe. Dans le même sens, j'ai évoqué le rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme paru en juillet dernier. Il a conduit le Conseil des droits de l'homme des Nations unies à instaurer une mission de vérification des faits sur place. Ces initiatives nous semblent de nature à démêler

également pour nous d'éviter, de manière concrète, que le régime n'ait les moyens de poursuivre sa répression et les atteintes aux droits de l'homme. En novembre 2017, à la suite des répressions de manifestations observées sur place en 2014 et 2017, l'Union européenne a mis en place un embargo sur les matériels de guerre et les équipements sensibles pouvant être utilisés pour la surveillance et la répression de la population vénézuélienne par le régime de Nicolás Maduro. Ces dispositions, vous l'imaginez- il n'est pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même -, sont bien sûr strictement appliquées par la France. La France a noté que le régime de Nicolás Maduro recourait à d'autres acteurs extérieurs pour maintenir son contrôle sur la population. Nous exhortons- je le fais très solennellement ici devant vous -l'ensemble des États à favoriser des négociations qui sont d'abord politiques.

des fonds : je tiens à le dire ici, nous maintenons un effort continu en ce sens. L'Union européenne a annoncé, le 27 septembre, de nouvelles sanctions individuelles à l'encontre de 7 membres du régime vénézuélien directement impliqués dans des atteintes aux droits de l'homme, ce qui porte à 25 les personnalités vénézuéliennes sanctionnées par l'Union. Les sanctions sont envisagées comme un mécanisme d'incitation aux négociations, elles peuvent donc être modulées selon l'évolution de la situation sur place. Ces sanctions individuelles prévoient un gel des avoirs des personnalités vénézuéliennes concernées, qu'une interdiction d'admission sur le territoire de l'Union européenne, et donc en France métropolitaine, comme dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Au vu des atteintes renouvelées aux droits de l'homme et de l'impasse politique, nous étudions de nouvelles possibilités de désignations individuelles avec nos partenaires européens. L'action de la France, saluée par nos interlocuteurs et vous-mêmes, conjugue donc l'appui aux négociations et la pression sur les autorités vénézuéliennes, au moyen de sanctions individuelles décidées avec nos partenaires européens. Je voulais, pour conclure, vous dire que, au fond, nous soutenons cette résolution sur son analyse de la situation et sur la nécessaire pression à exercer sur les autorités vénézuéliennes actuelles. Sur le point spécifique de la saisine de la Cour pénale internationale- et donc sur votre demande implicite que la France rejoigne les pays signataires du dossier en cours devant la CPI

alors qu'il risque d'être instrumentalisé et politisé, et qu'il constitue ainsi bien un préalable. Sans préjuger de ses conclusions, nous suivrons très attentivement son évolution. Cela ne nous empêche pas d'être attentifs aux travaux menés et de tirer, ensuite, toutes les conséquences quand les faits auront été établis et caractérisés par la CPI. J'espère ainsi, madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avoir pu répondre à vos interrogations. Je vous remercie à nouveau pour votre travail de vigilance sur ce sujet ô combien important en Amérique latine, mais aussi pour la